Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Gérard César, ancien sénateur de la Gironde. Nous honorons non seulement la mémoire du sénateur qu’il a été, de l’élu de terrain – il fut maire et conseiller général –, mais aussi et peut être avant tout le viticulteur, l’ardent défenseur du vin, patrimoine de la culture française. Ce viticulteur dans l’âme milita au sein du syndicalisme agricole et devint, au milieu des années 1960, président des Jeunes Agriculteurs de la Gironde. Il dirigea la belle cave coopérative de Rauzan. 1973, année durant laquelle il fut élu conseiller général du canton de Pujols, il devint suppléant de Robert Boulin. L’année suivante, il fut élu maire de Rauzan, fonction qu’il a exercée jusqu’en 2022.

Il siège alors au groupe du Rassemblement pour la République (RPR). Il est d’abord membre de la commission des affaires sociales, avant que nous ne nous retrouvions au sein de la commission des affaires économiques, dont il devient vice président en 2001.

attaché à cette terre qu’il arpentait entre les rangs de ses vignes, cette terre qui produit le Haut Mazières.

je vous remercie

président du groupe d’amitié France Maroc accompagné de sa vice présidente et de ses rapporteurs. La délégation est accompagnée par notre collègue Christian Cambon, président du groupe d’amitié France Maroc À l’invitation de ce groupe d’amitié, la délégation effectue une visite d’étude en France, qui l’aura conduite de Marseille et Toulon jusqu’à Paris ; elle s’est focalisée sur les questions de sécurité et de défense, en particulier en Méditerranée. Cette visite intervient alors que nous célébrons cette année le quatre vingtième anniversaire du débarquement en Provence, auquel les troupes marocaines ont éminemment contribué : souvenons nous, mes chers collègues, des dix mille Marocains morts pour la libération de notre pays Notre mémoire partagée rappelle la profondeur des liens tissés au fil de l’histoire entre la France et le Royaume du Maroc. Ce matin, j’ai eu plaisir à recevoir la délégation pour un entretien qui nous a permis d’identifier les prochaines étapes du rapprochement entre nos deux assemblées. Le dynamisme de notre coopération interparlementaire, qui doit tant au président Cambon, contribue éminemment à la relance, dans toutes ses dimensions, de la relation bilatérale franco marocaine, que nous appelons de nos vœux a également trouvé une expression forte dans le jumelage européen, achevé en mars 2023, dont le Sénat a été le chef de file, qui a marqué une collaboration intense entre nos chambres. En votre nom à tous, permettez moi de souhaiter à nos amis et collègues de la Chambre des conseillers du Maroc la plus cordiale bienvenue au Sénat français

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges

Avant d’aborder une série de questions dont certaines porteront sur la Nouvelle Calédonie, je souhaite appeler solennellement l’ensemble de la population calédonienne à la raison et au calme, comme viennent de le faire, dans un communiqué commun, les forces politiques calédoniennes, indépendantistes et non indépendantistes. Tout embrasement supplémentaire mettrait à mal le vivre ensemble et la construction du destin commun si cher aux signataires de l’accord de Nouméa. Il y a déjà eu trop de morts, ce n’est pas acceptable. Je tiens à rendre un hommage particulier aux forces de l’ordre, à leur courage et à leur engagement face au déchaînement de violence auquel elles font face depuis plusieurs jours ; le nombre de blessés en témoigne. J’ai une pensée particulière pour le gendarme qui lutte J’exprime également ma solidarité aux Calédoniens qui ont été victimes de ces débordements et exactions. Enfin, mes pensées vont aussi aux membres du personnel pénitentiaire qui, dans l’exercice de leur mission pour l’État de droit,

froidement et lâchement assassinés hier dans l’Eure. Ce drame absolu bouleverse évidemment l’administration pénitentiaire, dont je veux saluer l’engagement quotidien, au service de la République et des Français.

hier : la République. C’est sur nos lois qu’on a tiré, sur le respect de nos règles, sur des femmes et des hommes qui se battent, tous les jours, contre l’impunité.

pour les sanctionner le plus lourdement possible, est totale. Le ministre de l’intérieur a déployé des moyens absolument exceptionnels. L’enquête progresse ; évidemment, aucun moyen n’est économisé pour retrouver ces criminels. Je le redis : ils sont traqués, ils seront trouvés et ils paieront

tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour renforcer encore la protection que nous devons à nos agents pénitentiaires. Nous la leur devons, parce qu’eux mêmes protègent, chaque jour, notre République ! La parole

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin le décès de trois de nos compatriotes en Nouvelle Calédonie. Les habitants de l’archipel ont traversé une deuxième nuit de violences, plus terrible encore que la précédente. Là bas, le temps s’est arrêté des policiers et gendarmes ont été blessés, des gendarmeries prises d’assaut. Après vous, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, nous tenons ici à rendre un hommage appuyé au courage et à l’engagement des forces de l’ordre. Nos pensées émues vont à nos concitoyens calédoniens qui vivent dans l’angoisse, pris qu’ils sont au milieu des tirs, des incendies et des attaques à l’arme blanche. Nous sommes tous conscients que la violence doit cesser. Les premières victimes de ces violences sont les Calédoniens eux mêmes. Je tiens à saluer le courage des responsables politiques, loyalistes comme indépendantistes, qui ont appelé au calme. C’est ce sens des responsabilités qui doit s’imposer. L’accord de Nouméa a affirmé le destin commun de tous les citoyens de la Nouvelle Calédonie. Par trois fois, les Calédoniens ont eu à écrire ce destin. Par trois fois, ils ont choisi la République. Le projet de loi constitutionnelle que nous avons voté et que l’Assemblée nationale a adopté la nuit dernière est une étape nécessaire de ce processus, qui, depuis plus de trente ans, a toujours suivi la voie démocratique. Le temps est venu de panser nos blessures et d’ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune. Le Président de la République a tendu la main aux représentants calédoniens. La solution sera le dialogue. Nous avons tous la responsabilité de le rendre possible, car les violences n’apporteront pas de réponse pour le présent, elles ne panseront pas les blessures du passé et, plus grave encore, elles compromettront l’avenir de la population calédonienne et de sa jeunesse.

Ces violences ont provoqué des dégâts majeurs, blessé plusieurs centaines de personnes, parmi lesquels des dizaines de policiers et de gendarmes. Ces dernières heures, ajoutant au drame, plusieurs personnes sont décédées lors de ces violences. Je veux avoir une pensée pour elles elles et pour les Calédoniens qui veulent le retour au calme. Je veux le dire de nouveau devant vous, comme je l’ai fait hier à l’Assemblée nationale : aucune violence n’est justifiable ou tolérable ; la violence ne peut jamais être acceptée.

parviennent à garder leur sang froid, malgré les attaques, malgré parfois les tirs d’armes à feu. Ces policiers et ces gendarmes assument et tiennent courageusement leur rôle pour protéger les vies et permettre le retour au calme. Notre urgence, aujourd’hui, c’est le rétablissement de l’ordre et le retour du calme et de la sérénité. Ce matin, le Président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour aborder la situation en Nouvelle Calédonie. Des décisions fortes ont été prises.

de mars dernier, à une très large majorité, le Sénat a adopté le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Hier, l’Assemblée nationale l’a adopté à son tour. Ce texte s’inscrit dans la lignée du processus engagé depuis la décision souveraine des Calédoniens, affirmée par trois fois, lors de trois référendums, de demeurer dans la République. Le dégel du corps électoral est un enjeu démocratique ; je rappelle que le Conseil d’État nous a enjoint de prendre cette mesure. Il s’agit de permettre à des milliers de personnes nées en Nouvelle Calédonie, ou y résidant depuis de nombreuses années, de participer aux prochaines élections provinciales, qui sont des élections locales. Dans ce contexte, nous n’avons jamais cessé d’appeler au dialogue ; nous n’avons jamais cessé de créer les conditions du dialogue, en tendant la main à tous les acteurs, indépendantistes comme non indépendantistes. Nous gardons invariablement ce cap, le cap du dialogue. Nous cherchons, de nouveau, à créer les conditions d’un accord politique global. C’est pourquoi le Président de la République a annoncé qu’il ne convoquerait pas le Congrès immédiatement après l’adoption conforme du projet de loi constitutionnelle par l’Assemblée nationale. C’est pourquoi le Président de la République a écrit à l’ensemble des responsables calédoniens pour leur proposer de se réunir à Paris et de tenter, de nouveau, de trouver un consensus.

je veux d’abord exprimer tout mon soutien aux familles des agents décédés, ainsi que de ceux qui ont été gravement blessés, dans l’assaut ignoble et barbare d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure. Une telle violence n’est pas tolérable, justice doit être faite Cette attaque survient quelques semaines avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques dans notre pays. Ces Jeux sont une chance formidable pour la France, pour notre rayonnement et pour notre économie,

Nos policiers et nos gendarmes doivent en effet assurer le maintien de l’ordre public, malgré des émeutes de plus en plus violentes et récurrentes. Les forces de l’ordre sont également engagées dans la lutte contre la drogue, à travers des opérations « place nette » de grande ampleur. Elles doivent enfin continuer de protéger nos concitoyens contre la menace terroriste, portée au niveau d’alerte « urgence attentat ». Nous saluons le travail de ces femmes et de ces hommes. Plus que jamais, ils assurent une mission essentielle sans ménager leurs efforts. Dans un tel contexte, certains s’inquiètent de notre capacité à maintenir l’ordre : parviendrons nous à assurer la sécurité des jeux Olympiques sans fragiliser celle des territoires les plus reculés,

Les directeurs d’établissement dénoncent l’impact de l’inflation sur les charges d’exploitation, mais également la compensation incomplète des revalorisations salariales et l’évolution insuffisante des tarifs d’hébergement. La situation pousse ces responsables à chercher à faire des économies sur tout et sur tous

des 95 %. Ce n’est pas une question de volonté de la part des membres du personnel de ces établissements : dans ces conditions précaires, ils font preuve d’un dévouement que nous pouvons saluer. La question du financement de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale, relative à l’autonomie, reste au cœur du débat. doit faire l’objet de choix concrets, à la hauteur des besoins du secteur, qui devront permettre de ne plus faire peser sur les résidents ou leurs familles cette situation budgétaire intenable. Aussi, monsieur le Premier ministre, afin de garantir aux Ehpad les moyens d’assurer un accompagnement respectueux de la dignité des personnes âgées, quelle réforme de leur financement envisagez vous ? La parole

des femmes et des hommes qui, dans leur écrasante majorité, se donnent sans compter et s’engagent pour les autres ; je veux leur rendre hommage avec vous. Nous devons répondre aux défis des Ehpad,

Nous répondons présent pour rétablir la confiance dans ces établissements, avec un vaste plan de contrôle. Nous répondons présent aussi, évidemment, pour préserver leur viabilité. Tel est le sens du fonds d’urgence de 100 millions d’euros créé l’an dernier, ainsi que de l’augmentation inédite des dotations entre 2019 et 2023, : cela signifie 4 milliards d’euros de plus pour nos aînés, pour que le personnel des Ehpad soit mieux payé et plus nombreux. Malgré tout, je sais que des établissements connaissent toujours

la possibilité de définir deux tarifs d’hébergement différenciés en fonction des revenus. Ces mesures sont importantes, mais je pense, comme vous, que nous devons aller plus loin, notamment en faisant évoluer la gouvernance Mon gouvernement a donc proposé aux présidents de conseils départementaux une expérimentation qui verrait l’État financer la dépendance, comme le demandent les professionnels. Près d’un quart des départements s’y sont portés candidats, et je souhaite que le mouvement se poursuive. Par ailleurs,

et Républicain. Monsieur le Premier ministre, il est minuit à Nouméa et, à 17 000 kilomètres de Paris, la République vacille. La Nouvelle Calédonie s’embrase et renoue avec une histoire douloureuse de tensions et de violences, que je condamne. Trois personnes ont été tuées lors de la dernière nuit d’affrontements. C’est dramatique. Mes pensées vont aux familles endeuillées. Je veux aussi apporter tout mon soutien aux sapeurs pompiers et aux membres des forces de l’ordre déployés sur le terrain, qui ont à déplorer plus d’une centaine de blessés, parmi lesquels un gendarme se trouve entre la vie et la mort. L’ordre républicain doit être rétabli en Nouvelle Calédonie, dans les rues autant que dans les esprits. Pour cela, il faut naturellement une réponse sécuritaire, mais il faut aussi construire de justes équilibres pour parvenir à une désescalade de la crise. Le temps long est la condition d’un débat serein, sur l’archipel plus que nulle part ailleurs. Nous vous avons alerté en vain à maintes reprises. Le 7 mai encore, mon collègue député Boris Vallaud et moi même avons soumis nos propositions au Président de la République. Pour sortir de cette crise, il faut renouer avec la lucidité, l’humilité et l’impartialité qui prévalaient depuis 1988. Il faut créer immédiatement une mission de dialogue entre tous les partenaires calédoniens et l’État. Il faut annoncer que le Congrès ne sera pas convoqué. Il faut aboutir, sans ultimatum dans le temps, à un accord global tripartite dont vous devez être le garant, monsieur le Premier ministre. Vos appels au calme ont été totalement improductifs, car ce dossier ne devait pas quitter le bureau historique du Premier ministre. En conséquence, allez vous interrompre le processus constitutionnel ? Allez vous enfin vous engager personnellement ? Allez vous vous rendre en Nouvelle Calédonie ?

d’influences étrangères. Vous avez délibérément décidé de tourner le dos à une méthode éprouvée depuis 1988 par Michel Rocard, puis par Lionel Jospin.

votre rôle, c’est de prévenir les crises, non d’éteindre les incendies. Cécile Cukierman, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues,

que votre jusqu’au boutisme ainsi que celui du Président de la République ont plongé la Nouvelle Calédonie dans une crise profonde, marquée par la violence ? On dénombre déjà des centaines de blessés, notamment un gendarme, très grièvement blessé. Trois manifestants ont déjà été tués.

constitutionnelle qui remet en cause le processus de décolonisation issu de l’accord de Nouméa en actant le dégel du corps électoral. En faisant cela, vous avez fait vaciller la paix civile. Cessez donc vos éléments de langage ! Vous saviez qu’en poussant l’Assemblée nationale au vote du texte, véritable victoire à la Pyrrhus, vous fermiez la porte au dialogue.

la quasi totalité des groupes politiques au congrès de Nouvelle Calédonie. Il y a une heure, l’état d’urgence a été annoncé. Cette décision signe la faillite de votre politique. Je l’affirme solennellement c’est une faute démocratique lourde d’avoir recours à l’état d’urgence pour imposer un projet de loi, de surcroît un projet de loi constitutionnelle. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez, vous devez stopper cet engrenage. Allez vous retirer le projet de loi constitutionnelle

Parce que c’est un préalable à tout, parce que la violence ne peut jamais être justifiée ou acceptable. Pour le reste, j’ai déjà répondu à deux reprises, à MM. François Patriat Je rappelle le processus qui a été conduit ces dernières années par le Gouvernement, par Sébastien Lecornu, quand il était ministre des outre mer, par Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre mer. Il a permis

Monsieur le Premier ministre, le dialogue ne se décrète pas, pas plus qu’il ne s’impose. Il se construit dans le respect des forces en présence. Avec la méthode qui a été la vôtre, vous avez attisé le feu. Il est maintenant temps de l’éteindre et de reprendre sur de nouvelles bases la construction d’un avenir meilleur pour le peuple kanak comme pour la République française. La parole est à M. François Bonneau, pour le groupe Union Centriste.

confirmée par l’obtention du statut de candidat à l’Union européenne à la fin de 2023. Il s’agit là d’une avancée significative qui a renforcé les aspirations européennes de plus de 80 % de sa population. Cette dynamique se trouve aujourd’hui menacée. Nous observons avec une profonde préoccupation que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, dirigé par l’oligarque Bidzina Ivanichvili, adopte des lois qui tournent le dos aux valeurs et aux principes européens, malgré les avertissements répétés du Conseil de l’Europe et de la Commission de Venise. Plus particulièrement, le projet de loi sur la transparence de l’influence étrangère, évoquant étrangement la loi russe sur les agents étrangers, a suscité une vaste opposition au sein de la population et de très nombreuses manifestations à Tbilissi. Dans un contexte déjà alourdi par les tensions régionales liées à la guerre en Ukraine et la présence militaire russe dans les pays du Caucase du Sud, la Géorgie risque de se retrouver isolée à un moment très critique de son histoire moderne. La France a une relation historique avec la Géorgie, notamment marquée par l’accueil du gouvernement géorgien en exil de 1918 à 1921. Elle a joué un rôle clé dans la stabilisation post guerre russo géorgienne de 2008. Elle se doit aujourd’hui de prendre vigoureusement position. Nos engagements concernant l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie sont clairs, tout comme est manifeste notre soutien aux valeurs de démocratie et de liberté. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, franco géorgienne, incarne les liens entre nos deux pays et s’oppose avec beaucoup de courage aux caciques du parti en place. Monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments, comment la France prévoit elle de défendre nos intérêts stratégiques communs et de soutenir les Géorgiens dans leur aspiration européenne, malgré l’adoption de la loi controversée,

M. le ministre délégué chargé de l’Europe. Monsieur le sénateur François Bonneau, hier soir, comme depuis plusieurs semaines, le peuple géorgien s’est levé pour défendre la liberté et la démocratie, en bravant les violences et les milices, en brandissant le drapeau européen,

où l’Europe est tant décriée, dénigrée par les populistes et les nationalistes de tous bords, ce chant qui s’élève dans la nuit en Géorgie nous rappelle que l’Europe, c’est la liberté, que l’Europe, c’est la démocratie, que l’Europe, c’est l’espérance pour tant de peuples dans le monde.

ce message en Géorgie. Oui, la France déplore l’adoption de ce projet de loi, qui discrédite les ONG et les médias indépendants. La France condamne les violences contre les manifestations et appelle les autorités géorgiennes à faire respecter le droit de manifester pacifiquement et la liberté des médias. Oui, la France se tient aux côtés de la Géorgie dans son chemin vers l’Union européenne, qui est le seul auquel son peuple aspire. aspire. Chacun le sait ici, rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. La parole est à Mme Anne Souyris, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. Mme la ministre de la culture. Dimanche dernier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France appelaient à la grève, pour la liberté d’expression. Leur inquiétude est justifiée par une suite d’événements troublants, dans un contexte de montée de l’extrême droite, de politiques liberticides et de répression des manifestations, notamment étudiantes, au sein même de nos universités, dans notre pays et en Europe. D’abord, D’abord, l’humoriste Guillaume Meurice est suspendu par la direction de Radio France pour des propos tenus à l’antenne. S’ils interrogent, ces propos n’ont pas fait l’objet d’une condamnation par la justice – au contraire, la plainte a été classée sans suite. Ensuite, Mme Dati présente un projet de réforme de l’audiovisuel public, une sorte de « fusion acquisition » des médias publics. Lundi

sur l’environnement qui n’ont probablement pas beaucoup d’intérêt pour certains… Après tout, « qui aurait pu prédire la crise climatique ? » Je ne vous le demanderai pas ! Qui aurait pu prédire la crise

quand ils sont libres de s’exprimer. Madame la ministre, comment allez vous garantir le pluralisme et la liberté d’expression des médias publics, donc la démocratie elle même, avec cette réforme ? La

l’égard de l’information. Dans ce cadre, un projet de loi a été présenté, débattu et voté hier en commission à l’Assemblée nationale. Ce texte ne vient pas de nulle part, il s’inspire directement de travaux parlementaires,

S’il y a un risque, il vient de certains de vos alliés à l’Assemblée nationale, qui, pas plus tard qu’hier, appelaient à supprimer les éditorialistes et à menacer la liberté d’opinion. Charité bien ordonnée commence par soi même La parole est à M. Étienne Blanc, pour le groupe Les Républicains.

s’élève à 117 millions d’euros. Autant vous dire, monsieur le Premier ministre, que cette différence est absolument considérable.

du système de narcotrafic en France. Qui plus est, dans une République qui connaît des problèmes pour faire face au fonctionnement de sa justice, dont la police et la douane nous pouvons trouver là un gisement de ressources absolument considérable permettant de répondre aux besoins des services. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple

et le rappeler, à la suite du Premier ministre : au travers de ces agents de la pénitentiaire, c’est bien la République entière qui est gravement attaquée. Monsieur le sénateur Blanc,

J’y arrive. … et la violence de ces crimes inouïs conduit celui ci à adopter des mesures radicales contre le crime organisé. Dès le mois dernier, le garde des sceaux a annoncé des mesures fortes création d’un parquet national anticriminalité, cour d’assises spécialement composée pour les règlements de compte, statut du repenti, nouveau crime d’association de malfaiteurs. Monsieur le sénateur, à l’automne prochain, un projet de loi spécifique sera présenté.

Madame la ministre, votre absence de réponse est révélatrice de l’ampleur du désastre. La parole est à M. Georges Naturel, pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, depuis trois jours, je suis en lien étroit avec nos compatriotes calédoniens, soumis à la violence et à la peur, dans une situation insurrectionnelle et un chaos urbain. Vous connaissez le triste bilan. Il ne fait que s’alourdir. On dénombre déjà quatre morts.

les Calédoniens qui ont vu leurs biens ravagés et partir en fumée et qui sont reclus dans l’angoisse et la crainte, sans céder aux provocations.

tout l’objet de ma question. Comment comptez vous renouer les fils du dialogue dans le dossier calédonien ? Reprendrez vous personnellement le dossier ? Quels acteurs calédoniens participeront aux discussions annoncées à Paris ?

: après une nuit de protection dans un endroit particulièrement dangereux, où les tirs ont été effectués à balles réelles, des « vieux », comme l’on dit chez vous en Nouvelle Calédonie, sont venus parler aux gendarmes, il a alors retiré son casque, s’est fait tirer dessus et a reçu Depuis trois jours, alors que c’est la démocratie que nous rétablissons en Nouvelle Calédonie, conformément à la volonté du peuple calédonien qui s’est exprimée par trois fois, des centaines de policiers et de gendarmes sont blessés, leurs familles terrorisées.

au Parlement, des réunions se tenaient et je salue, comme l’ont fait le président du Sénat et le Président de la République, le communiqué commun de toutes les forces politiques. Reste qu’il ne faut pas confondre la pression politique, les manifestations et les contestations avec la violence, les tirs à balles réelles et les personnes qui pillent, qui tuent et qui en veulent à la République. Oui au dialogue, comme l’a dit le Premier ministre, autant qu’il le faudra, où il le faudra, avec qui il le faudra, mais jamais la République ne doit trembler devant les kalachnikovs. Merci

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur et des outre mer. Le drame qui s’est produit hier dans l’Eure a profondément ému la représentation nationale. Je veux exprimer au nom de mon groupe nos sincères condoléances aux familles et aux proches des agents blessés ou sauvagement assassinés.

de ce rapport, le Sénat appelle à « un nécessaire sursaut [pour] sortir du piège du narcotrafic ». Pourtant, monsieur le ministre, vous avez réitéré ce matin votre volonté d’attaquer le fléau par le bas. Nous pensons au contraire qu’il faut frapper les réseaux au portefeuille et à la tête. Monsieur le ministre, allez vous répondre à l’appel unanime du Sénat ?

faire des saisies et attaquer les consommateurs, mais personne ne doute un seul instant que le sénateur Blanc et vous même ayez raison : la confiscation doit être générale, l’argent du crime doit être confisqué et nous devons faire cent fois plus que ce que nous faisons collectivement.

Aux Pays Bas, en Belgique, on assassine des journalistes et des avocats et on assassine peut être putativement des hommes et des femmes politiques. En Amérique du Sud, la production de stupéfiants a été multipliée par cent parce que les États Unis se sont désintéressés

Monsieur le ministre, l’écart est grand entre le discours que vous tenez devant nous et les actes du Gouvernement. Vous affirmez que la drogue est la plus grande menace sécuritaire que notre pays et le monde vont connaître. Nous partageons cet avis, mais nous estimons que votre réponse n’est pas à la hauteur de la menace. Sur le terrorisme, nous sommes en ordre de bataille. Sur le narcotrafic, nous avançons en ordre dispersé. Corruption, outre mer, blanchiment, sécurité des ports, prison, procédure pénale, coopération internationale, magistrats et policiers en demande de moyens : tous les chantiers sont ouverts. Le Sénat propose la création

La parole est à Mme Catherine Belrhiti, pour le groupe Les Républicains. de la jeunesse. Madame la ministre, vous avez récemment reconnu les difficultés de recrutement des enseignants dans certaines académies pour la rentrée 2024. Les premiers résultats des écrits du concours de recrutement des professeurs des écoles affichent ainsi un ratio de candidats par poste largement inférieur aux précédentes décennies, et ce avant même les résultats définitifs. à ce constat, vous répondez chaque année par le recrutement de nouveaux contractuels, dans des conditions de formation loin d’être adaptées. La volonté gouvernementale de passer le concours de recrutement à bac+3 est une réponse bien insuffisante face à la gravité de la situation. Insérer nos futurs enseignants dans leur milieu professionnel selon les modalités actuelles ne conduira qu’à les exposer à plusieurs problèmes systémiques de l’éducation nationale la rémunération, le déroulement des carrières, la mobilité et le manque de reconnaissance. Qui aujourd’hui souhaiterait gagner 1,1 fois le Smic en début de carrière après cinq années d’études ? De plus, le système de gestion des ressources humaines, qui ne fonctionne qu’à l’ancienneté, conduit à envoyer de jeunes professeurs loin de chez eux, dans les territoires réputés les plus difficiles. Cela revient souvent à leur demander de sacrifier leur projet de vie. Madame la ministre, quand le Gouvernement se décidera t il enfin à mettre en place un pacte qui rendra à la profession son attractivité et offrira à la jeunesse de ce pays un avenir ?

de modifier la formation initiale de nos personnels. Nous mettons en place – c’est véritablement une réforme structurante et enthousiasmante – une formation d’excellence.

Vous traitez le problème d’attractivité par de petites réformes mises bout à bout, alors que nous avons besoin de repenser la profession en prévoyant un véritable plan d’insertion des jeunes professeurs. Par exemple, la régionalisation des concours semble aujourd’hui une étape indispensable. Madame la ministre, sans une réforme d’ampleur, sans ce nouveau pacte fondateur, la contractualisation de l’éducation nationale est inexorable. Soyez en assurée, les professeurs qui ne s’épanouissent pas dans leur métier ne seront pas en mesure de former les têtes bien faites de demain ! La parole est à M. Guislain Cambier, pour le groupe Union Centriste.

renforcer la formation et la professionnalisation des médecins généralistes afin de faciliter et de sécuriser leur installation ; d’autre part, répondre aux besoins de santé croissants de la population, en particulier dans les territoires plus isolés et moins dotés en ressources médicales. de beaux objectifs, mais rien n’est prêt ! Dans nos territoires, les élus, les médecins, les formateurs et les étudiants nous alertent sur l’urgence de publier les textes réglementaires. Les futurs généralistes concernés ont en effet débuté leur internat en 2023. Votre prédécesseur avait acté oralement plusieurs arbitrages qui ont engagé la parole de l’État auprès des étudiants, des professionnels et de la population. Mais, à ce jour, aucun texte relatif aux questions évoquées n’a été publié. De ce fait, dans mon département, le Nord, beaucoup de praticiens nous disent qu’ils n’ont pas la place dans leur cabinet pour recevoir les 250 docteurs juniors programmés par an.

et orienter nos médecins vers nos territoires. Mais mettre à disposition de nouveaux locaux, des logements et, éventuellement, les construire nécessite un calendrier précis. Monsieur le ministre, dans quels locaux les docteurs juniors exerceront ils ? Sous quelle autorité ? Quelle sera leur formation, et celle des maîtres de stage ? de leur rémunération et de leur logement ? La

la médecine générale est essentielle à l’avenir de notre système de santé. C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité envoyer un signal fort d’attractivité et de reconnaissance – c’est un terme que vous avez employé –, afin que les jeunes soient de plus en plus nombreux à choisir cette voie et à s’installer dans nos territoires. Conformément aux engagements du Président de la République, mes prédécesseurs, en lien avec Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont engagé une réforme ajoutant une quatrième année

La nouvelle maquette de formation du diplôme d’études spécialisées de médecine générale a été publiée l’an dernier. Elle a suscité des interrogations de la part des internes et de nombreux acteurs. Aussi ai je demandé à des personnalités qualifiées de poursuivre la concertation nécessaire à l’identification des conditions de succès.

Un accord pourrait même être prochainement adopté lors de la 77 Assemblée mondiale de la santé, qui se tiendra dans quelques jours. La réponse aux pandémies suppose que tous les pays soient intégrés aux dispositifs de l’OMS, sans exclusion et sans réserve. À plusieurs reprises, la France s’est déclarée favorable à la participation de Taïwan au sein d’instances de l’OMS, reconnaissant son expertise médicale, par la voix de M. Le Drian en 2021 ou celle de Mme Colonna en 2023. Cependant, il faut constater que, à part quelques réunions chichement autorisées par an, Taïwan ne peut pas s’impliquer dans des mécanismes comme le système mondial de surveillance de la grippe et de riposte ou le réseau mondial de vérification sanitaire numérique. Taïwan n’est ainsi pas en mesure de délivrer et de vérifier des documents de certification numérisée conformes aux normes internationales. En cas de nouvelle pandémie, cela créerait des difficultés pour les Taïwanais travaillant à l’étranger, mais aussi pour tous les étrangers vivant à Taïwan, dont plusieurs milliers de Français. Cette exclusion de Taïwan est contraire aux objectifs de l’OMS, empêche la lutte contre les virus et nuit à la santé de toutes les populations. Taïwan doit pouvoir participer pleinement aux activités de l’OMS. La lutte contre les pandémies ne saurait être sacrifiée du fait de pressions mesquines. Je vous demande donc de prendre des mesures concrètes en faveur de Taïwan. Pourquoi faire preuve de lenteur alors qu’on sait visiblement dérouler le tapis rouge pour certains ? Qu’attendez vous pour que Taïwan soit pleinement intégrée à l’OMS ? Pourquoi tant d’hésitations ? La santé publique mondiale et la santé des Français n’attendent pas

je connais votre intérêt pour le sujet, vous qui êtes vice présidente du groupe d’échanges et d’études Sénat Taïwan, présidé par Jean Baptiste Lemoyne. Comme chaque année, la question de la participation de Taïwan à l’Assemblée mondiale de la santé est soulevée. La position de la France est connue et constante : il n’y a qu’une seule Chine. Nous soutenons cependant, dans le respect de la politique d’une seule Chine, la participation de Taïwan aux travaux des organisations internationales lorsque leur statut le permet et lorsque c’est dans l’intérêt collectif. Notre position sur ce point n’a pas changé ; elle a d’ailleurs été exprimée devant cette assemblée à plusieurs reprises. Je l’ai indiqué, la France s’en tient depuis 1964 à sa politique constante d’une seule Chine et n’a pas de relations diplomatiques avec Taïwan. Cela n’empêche en aucun cas le développement de coopérations riches avec Taïwan dans de très nombreux domaines. C’est dans cette perspective que nous appelons l’OMS, dans le respect de ses statuts, à inclure davantage Taïwan dans ses travaux, notamment à l’occasion de l’Assemblée mondiale de la santé, qui aura lieu

merci beaucoup de votre question ! Je crois que nul ici ne peut accuser la France, le Président de la République ou le Gouvernement de manquer de fermeté à l’égard de la Russie de Vladimir Poutine. Dès les premiers jours de l’offensive russe en Ukraine, c’est la France qui a pris l’initiative de proposer le premier des quatorze paquets de sanctions ayant visé les intérêts russes et gelé les avoirs, avoirs dont les revenus seront désormais utilisés pour financer le soutien militaire à l’Ukraine.

! Que faisait il là bas ? Notre ambassadeur de France en Russie, en poste depuis quatre ans, exerce ses responsabilités dans des conditions extrêmement difficiles et sous la pression permanente du pouvoir russe.

L’attractivité de notre pays repose en grande partie sur des dispositifs fiscaux, comme le crédit d’impôt recherche, qui fait de la France une terre de recherche avant d’être une terre de production.

Leur incidence réelle en matière d’emploi suscite donc des interrogations. Monsieur le ministre, pouvez vous nous assurer que les projets d’investissements qu’accueille la France auront un effet réel et durable en termes d’emplois et de valeur ajoutée ?

Mais je m’en réjouis, croyez le bien, monsieur le ministre ! Simplement, il y a les annonces et il y a les chiffres. Or les chiffres sont têtus. Selon le dernier baromètre Ernst & Young, la rentabilité des investissements étrangers en termes d’emplois est plus faible chez nous que chez nos voisins.

Ils sont accompagnés d’une trentaine d’académiciens et de chercheurs, ainsi que des députés et sénateurs membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, présidé par le sénateur Stéphane Leur présence s’inscrit dans le cadre d’un partenariat noué par l’Office avec les Académies

elle induit pour la prise en charge du recyclage des produits en fin de vie des tarifs discriminants, jusqu’à six à vingt fois plus élevés que ceux qui sont appliqués, par exemple, aux structures en béton ou en acier.

Imposer de tels surcoûts au bois, matériau renouvelable de construction et de décarbonation, alors que les enjeux de la planification écologique et de la construction de logements sont devant nous, est un non sens. En fait, monsieur le ministre, c’est le barème de cette REP qui pose problème. Il n’est pas adapté aux réalités et il doit être revu. Il ne tient aucun compte du cycle de vie vertueux et du profil écologique des produits en bois. Qui plus est, il ignore que le bois de déconstruction est déjà aujourd’hui largement trié, valorisé, valorisé, réutilisé dans la production de panneaux, de palettes ou en biomasse énergie. C’est donc une économie circulaire vertueuse qui est en place, mais elle n’est pas prise en compte

–, nous allons moduler les niveaux de financement des matériaux en fonction de la réalité de la collecte et du recyclage. Compte tenu de ce que vous décrivez dans la filière bois, le décret, qui devrait être publié, je l’ai dit, au plus tard à la fin du mois de juin, permettra de remettre de l’équité

La séance est reprise. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection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

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est avant tout un texte de justice et d’humanité. C’est un texte d’humanité, parce que l’enjeu est de ne pas ajouter de la fragilité à la fragilité. Sans encadrement, les frais bancaires au moment des successions viennent ajouter à la perte d’un proche l’inquiétude face aux coûts à supporter. de justice, parce que ces frais peuvent être excessifs. Tel est le sens de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. Je veux saluer le travail qui a permis sa construction, tout comme l’engagement des parlementaires, au premier rang desquels la députée Christine Pires Beaune et le sénateur Hervé Maurey je connais leur investissement à tous les deux sur le sujet. Mesdames, messieurs les sénateurs, dès le dépôt de ce texte, le Gouvernement et la majorité ont été à vos côtés pour lui permettre d’aboutir. Olivia Grégoire avait eu l’occasion de le rappeler devant l’Assemblée nationale : le Gouvernement agit depuis 2017 pour limiter les frais bancaires des plus fragiles. En 2019, le Gouvernement a élargi les critères permettant d’être reconnu comme « fragile », situation qui donne le droit à un plafonnement des frais bancaires. Depuis lors, près de 700 000 Français supplémentaires bénéficient de ce plafonnement.

Au delà de la lutte inlassable que nous menons contre les fraudeurs,… Bravo ! … il est aussi de notre responsabilité de protéger ceux qui en sont victimes. Le texte qui nous réunit aujourd’hui sur les frais de clôture du compte d’un défunt est l’aboutissement d’un engagement, d’un engagement, celui de Bruno Le Maire, qui avait permis, dès 2021, la réduction des frais appliqués par certaines banques. Cet engagement méritait d’être traduit dans la loi pour devenir une règle uniforme, appliquée par tous. C’est l’objet de ce texte, que le travail parlementaire mené en particulier par le rapporteur au sein de la commission des finances du Sénat a permis de modifier et d’enrichir. Pour prévenir toute confusion et garantir le respect des exigences constitutionnelles en matière d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, la structure de l’article 1 a été modifiée afin de clarifier les différents cas de gratuité. Trois cas ont ainsi été définis, ciblant à la fois les clients les plus modestes et les successions les plus simples. Ils permettront de couvrir entre 30 % et 40 % de la population, soit une part importante des Français. En particulier, il n’y aura plus de frais lorsque l’héritier justifiera de sa qualité d’héritier dans les conditions de la procédure de clôture des comptes simplifiée ; lorsque le montant total des soldes des comptes sera inférieur à un seuil fixé à 5 000 euros ; et enfin lorsque le détenteur des comptes est mineur à la date du décès. Ce dernier point est particulièrement important, car, si tous les deuils sont difficiles, il est d’autant plus insupportable de s’acquitter de frais bancaires lorsque l’on vient de perdre son enfant. Pour autant, ce texte ne remet pas en cause la réalité des coûts auxquels les banques doivent faire face. Avant la clôture des comptes d’un défunt, les banques engagent des opérations préalables à la succession. Par exemple, elles accompagnent la famille du défunt dans l’obtention des pièces justificatives ; elles vérifient l’authenticité de l’acte de décès ; elles peuvent s’occuper du gel des avoirs et de leur déclaration à l’administration fiscale, des échanges avec le notaire, de la désolidarisation éventuelle des comptes joints ou encore du transfert des fonds aux héritiers selon les ordres du notaire. Il faut aussi tenir compte de la matérialité des coûts administratifs effectivement supportés par les banques pour identifier sans erreur les ayants droit du défunt avant de leur verser les fonds. C’est pourquoi la gratuité est ciblée. Dans les cas non couverts par cette gratuité et en cohérence avec la mesure portée par le rapporteur Hervé Maurey et adoptée par le Sénat en 2023, la commission des finances a par ailleurs prévu un barème pour le plafonnement des frais, qui sera déterminé par décret d’application. Celui ci ne pourra pas dépasser 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne. De plus, les frais prélevés par les établissements de paiement, dont les offres attirent un nombre croissant de clients, ont été inclus dans le dispositif. En complément, les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont expressément habilités à contrôler le respect de ces nouvelles règles d’application. Ce texte complet et équilibré est donc l’aboutissement d’un travail riche et transpartisan pour mieux accompagner les Français dans les moments difficiles qu’ils traversent. Mesdames, messieurs les sénateurs, réduire et encadrer les frais bancaires liés au décès d’un être cher, c’est bien le sens du texte que le Gouvernement soutiendra et qui nous rassemble, au delà des clivages, autour d’un impératif : celui de plus d’humanité face au deuil, que chacun d’entre nous est amené, un jour ou l’autre, à affronter.

parmi les différents types de frais bancaires, les frais appliqués dans le cadre des opérations de succession se distinguent par leur disparité, leur coût élevé et leur manque de transparence. Ces frais représenteraient selon les estimations entre 125 millions d’euros et 200 millions d’euros par an, soit environ 1 % de l’ensemble des frais bancaires prélevés en France. Si ce montant peut sembler marginal au regard de l’activité des banques, les sommes prélevées pour une succession peuvent être significatives, notamment pour les successions les plus modestes. Selon une étude de l’UFC Que Choisir, les frais bancaires acquittés par les héritiers pour une succession de 20 000 euros peuvent varier de 80 euros à 527,50 euros. Avec une moyenne de 291 euros en 2023, en hausse de 25 % par rapport à 2021 et de 50 % par rapport à 2012, les frais bancaires facturés en France au titre des opérations liées aux successions seraient trois fois supérieurs à ceux qui sont pratiqués en Belgique et en Italie, et même quatre fois plus élevés qu’en Espagne. Le cas de parents qui se sont vu réclamer 138 euros pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans, décédé, a créé une vive émotion et suscité un certain nombre de réactions comme d’initiatives parlementaires. C’est ainsi que dès le mois de novembre 2021, j’ai interrogé le ministre Bruno Le Maire sur les mesures qu’il comptait prendre pour remédier aux difficultés observées. Dans sa réponse de janvier 2022, le ministre assurait que le Gouvernement demeurait « à ce titre déterminé à ce qu’une solution soit rapidement dégagée dans le cadre des instances de concertation de place ». Ne voyant pas le sujet évoluer du côté du Gouvernement, j’ai déposé une proposition de loi visant à encadrer les frais bancaires sur succession et prévoyant que ces frais soient « en rapport avec les coûts réellement supportés » par les établissements teneurs de comptes. Dans un courrier de septembre 2022, le ministre Bruno Le Maire, que j’avais de nouveau sollicité, renouvelait son engagement de faire évoluer les pratiques des banques « d’ici au début de l’automne ». Nous étions alors en 2022. En l’absence d’avancée, le Sénat s’est saisi de ce sujet en janvier 2023 lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants de nos collègues Jean François Husson et Albéric de Montgolfier. Notre assemblée avait alors adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques, respectivement déposés par Vanina Paoli Gagin et par moi même. Ces deux amendements prévoyaient la gratuité pour les comptes inférieurs à 5 000 euros bénéficiant de la procédure de clôture simplifiée et instituaient, pour les autres cas, un plafonnement à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement. Pour justifier l’avis défavorable du Gouvernement, le ministre Jean Noël Barrot promettait en séance la conclusion d’un accord de place « dans un délai d’un mois ». Nous étions, je le rappelle, Je tiens à souligner le caractère illusoire de l’accord de place longtemps recherché par le Gouvernement et je m’en étonne. En effet, les représentants des acteurs bancaires m’ont indiqué en audition qu’un tel accord n’avait jamais été envisagé, était manifestement contraire au droit de la concurrence. Celui ci prohibe en effet les ententes sur les prix, sous peine de sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires des activités concernées. Je suis donc assez surpris, rétrospectivement, de la position du Gouvernement. Aussi, je me réjouis que la députée Christine Pires Beaune ait pris l’initiative de porter de nouveau cette question devant le Parlement au travers de la présente proposition de loi. Je tiens à saluer son engagement et le fait qu’elle se soit toujours référée aux travaux du Sénat, tant dans ses interventions à l’Assemblée nationale que dans les médias. Je me réjouis – et l’en félicite – qu’elle ait réussi à convaincre enfin le Gouvernement de remédier à cette situation et de soutenir cette proposition de loi. Reconnaissant la grande qualité des travaux réalisés par la rapporteure à l’Assemblée nationale, j’ai abordé la présente proposition de loi avec l’objectif d’un vote conforme. En effet, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le dispositif proposé est tout à fait équilibré. Il prévoit trois cas de gratuité répondant aux situations les plus problématiques : en premier lieu, les successions les plus simples, c’est à dire lorsque l’héritier justifie de sa qualité auprès de l’établissement de crédit teneur des comptes par la production d’un acte de notoriété ou d’une ou d’une attestation signée par l’ensemble des héritiers ; en deuxième lieu, lorsque le montant total des soldes des comptes est inférieur au seuil de 5 000 euros, qui concerne les successions les plus modestes et 30 % de la population ; en troisième lieu, enfin, lorsque le détenteur des comptes était mineur à la date du décès. Dans les autres cas, les opérations liées à la succession pourront donner lieu à un prélèvement de frais, dont il reviendra au décret d’application de définir le barème. Cependant, à la suite de mes auditions et de mes entretiens avec vos services, monsieur le ministre – je les remercie de leur disponibilité et de leur fructueuse collaboration –, il m’est apparu nécessaire de conforter l’intelligibilité et la validité juridique de l’encadrement législatif envisagé. La commission des finances a donc procédé à une réécriture globale de l’article 1, qui porte le dispositif d’encadrement proposé. Concernant la gratuité relative aux successions modestes,

ce montant était de 5 909,95 euros. En ce qui concerne le cas de gratuité relatif aux successions les plus simples, une référence à l’absence de « complexité manifeste » a été introduite par la commission. Ces critères devront être détaillés par le décret d’application. Néanmoins, la notion de « complexité manifeste », inédite au sein du code monétaire et financier, reste sujette à interprétation. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement visant J’ai également déposé un amendement, rédactionnel, afin d’améliorer encore l’intelligibilité du dispositif, ainsi qu’un autre, visant à sécuriser sa date d’entrée en vigueur. La commission a par ailleurs élargi le champ d’application de l’encadrement, afin d’inclure les établissements de paiement tels que Nickel et Revolut, qui attirent un nombre croissant de consommateurs, notamment parmi les plus jeunes. De même, en vue d’assurer le contrôle de la mise en œuvre des nouvelles règles, la commission a prévu l’habilitation expresse des agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au delà de ces modifications qui viennent compléter et préciser utilement le texte de l’Assemblée nationale, nous avons souhaité reprendre le dispositif adopté en 2023 par le Sénat, qui prévoit que le barème tarifaire qui sera fixé par décret respecte un plafond de 1 % du montant total des soldes des comptes et produits d’épargne du défunt. Je précise – et j’insiste sur ce point – qu’il s’agit d’un maximum il n’est nullement question de prévoir que ce pourcentage s’applique à l’ensemble ni même à la majorité des successions non couvertes par la gratuité. De surcroît, ce premier plafond de 1 % sera complété par un second plafond en valeur, qui sera déterminé par le pouvoir réglementaire. Ainsi, l’application de ce double plafonnement ne saurait en aucun cas conduire à ce que les frais prélevés soient supérieurs aux niveaux actuels. Il appartiendra au Gouvernement d’y veiller scrupuleusement en prévoyant un barème dégressif en fonction du montant total des soldes, et ce, quels que soient les arguments, et même – j’ose le mot – les pressions des établissements bancaires. Rappelons que, pour une succession de 20 000 euros, le montant moyen de frais prélevés est aujourd’hui de 291 euros. Soulignons également que le patrimoine financier liquide transmis dans le cadre d’une succession représente, en moyenne, environ 10 000 euros. Dans le cadre du dispositif proposé, près de 50 % de nos concitoyens acquitteraient ainsi, au maximum, 100 euros de frais. Globalement, près de 80 % de nos concitoyens, je le souligne, acquitteront au maximum 200 euros de frais. Ce double plafonnement, en pourcentage et en valeur, constitue donc une protection majeure pour les consommateurs. Je ne m’attarderai pas sur les deux autres articles de cette proposition de loi, qui ne présentent pas de difficulté particulière. L’article 1 prévoit l’application du dispositif à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article 2 porte sur la remise d’un rapport destiné à évaluer l’impact des nouvelles règles un an après la publication du décret d’application. La commission des finances vous propose donc un dispositif équilibré et clarifié, pour enfin encadrer au niveau législatif les frais prélevés par les banques et par les établissements de paiement dans le cadre des opérations liées aux successions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les lois s’accumulent, mais la domination des banques demeure. Sans aucun doute, les frais bancaires constituent un élément de cette domination, faisant des citoyens des « sujets bancaires », si vous me permettez cette expression.

Pourtant, comme l’indique la rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale, la Fédération bancaire française a affirmé qu’il n’avait jamais été question de trouver un accord de place sur ce sujet. Comme souvent, il reste la loi pour imposer des choix de société, remédier à des injustices, lutter contre des dérives. La demande sociale est forte, l’aspiration à la protection face à une finance agressive est grande. Même s’ils ne représentaient que 1 % des frais totaux pratiqués, même une courbe exponentielle, trois fois supérieure à l’inflation. D’après l’association UFC Que Choisir, dont nous saluons la mobilisation, ces frais ont explosé pour atteindre en moyenne 291 euros à la fin de 2023, soit une hausse de 25 % en deux ans. Nous aurions pu les interdire purement et simplement, en dépit de ce qu’affirment la Fédération bancaire française et, parfois, certains de nos collègues de droite, qui légitiment le coût des opérations qui incombent aux banques dans le cadre de successions dites complexes. Étonnant, alors que certaines banques pratiquent d’ores et déjà la gratuité et que le Crédit mutuel, pour ne pas le citer, fait de même dans la limite de 10 000 euros ! Aucuns frais ne sont pourtant corrélés à l’encours du compte en banque. Le plafonnement à 1 % des frais du compte est alors purement artificiel et nous ne soutenons pas cette disposition. La commission des finances du Sénat aurait pu choisir un vote conforme. Le choix a été fait de modifier cette proposition de loi à la marge, notamment en y ajoutant la gratuité sans limite de montant pour les opérations dites simples. Mais nous ne sommes pas convaincus, toutefois, que cette avancée justifie de renoncer à un vote dans les mêmes termes. Je renouvelle notre demande d’une loi cadre. Ne nous limitons pas à des propositions de loi à la découpe. En effet, les frais pour incidents de paiement rapportent 6,5 milliards d’euros aux banques chaque année.

décorrélés du coût des opérations. Voilà la réalité sombre, anarchique ou presque, du marché des comptes de dépôt et des livrets, sans parler des produits financiarisés, pour lesquels règne la plus grande opacité. Cette

Je salue, une nouvelle fois, le rôle de lanceur d’alerte des associations de consommateurs. Dès 2021, l’UFC Que Choisir a dénoncé les pratiques abusives des banques françaises dans l’application de frais spécifiques aux successions : ceux ci n’ont pas de lien avec les coûts réels supportés par les établissements bancaires et pénalisent davantage les petites successions. Les opérations bancaires de contrôle des successions sont administratives : vérification de l’authenticité de l’acte de décès, gel des avoirs, déclaration à l’administration fiscale, échanges avec le notaire, désolidarisation des comptes joints, transfert des fonds aux héritiers sur ordre notarial, Les tarifs s’avèrent très disparates d’un établissement à l’autre, y compris au sein d’un même groupe, sans justification, et leur caractère immoral est, à juste titre, dénoncé. À l’heure de la dématérialisation des opérations financières, comment justifier de facturer 80 euros pour un virement final de succession, alors qu’un simple virement est gratuit du vivant de l’intéressé ? L’association de défense des consommateurs a relevé des frais bancaires de succession atteignant 200 euros, alors que le solde du compte bancaire était de 500 euros. Les héritiers se retrouvent pieds et poings liés face à des conditions contractuelles opaques, abusives et disproportionnées.

Il y a deux ans, le Gouvernement avait demandé au secteur bancaire de s’autoréguler, mais sans résultat. Face à cet immobilisme, il est urgent de mettre un terme à ces abus. Le texte que nous examinons a été adopté à l’Assemblée nationale, à l’unanimité, le 29 février dernier. Sa version initiale comportait un article unique, qui renvoyait les modalités de calcul des

Les disparitions prématurées sont un drame pour les familles. Beaucoup de jeunes de moins de 30 ans décèdent brutalement, parfois à la suite d’un accident de voiture ou, souvent, malheureusement, d’un suicide.

est le fruit d’une volonté transpartisane de remédier à une injustice financière, celle des prélèvements de frais disproportionnés par les établissements bancaires lors des successions. Je souhaite tout d’abord saluer le travail et la pugnacité de la députée socialiste Christine Pires Beaune, rapporteure de ce texte à l’Assemblée nationale, qui l’a fait adopter à l’unanimité en février dernier. J’espère que ce sera également le cas ici.

a été régulièrement évoqué dans les médias ces dernières années. En effet, certains prélèvements de frais ont pu parfois manquer de cette empathie et de cette humanité tant nécessaires dans ces moments. Je pense notamment au cas, particulièrement médiatisé, de Léo, enfant originaire de Gironde, décédé d’un cancer en 2021 à l’âge de 9 ans, dont les parents se sont vu prélever 138 euros de frais bancaires pour la clôture de son livret A.

2024, les frais bancaires sur succession sont, en France, en moyenne, de 303 euros. Ils ont augmenté de plus de 25 % depuis 2021, ce qui illustre leur déconnexion avec les réalités économiques.

Par exemple, dans l’une des banques de Nouvelle Calédonie, les frais prélevés sont de 191 euros pour l’ouverture d’un dossier de succession, auxquels s’ajoutent 115 euros par an et par compte concerné.

proche. Certaines prestations qui ne sont pas facturées du vivant du client, tel le transfert des fonds vers un autre établissement, deviennent onéreuses lorsqu’il s’agit de comptes du défunt. En effet, si la clôture du compte est gratuite au titre de l’article L. 312–1–7 d’autres opérations bancaires liées à la succession peuvent faire l’objet de frais dès lors que la somme des encours est supérieure à 5 000 euros. C’est pour cela qu’il est important de poursuivre le travail d’encadrement des frais bancaires pour les plus fragiles et les publics les plus en souffrance.

plus de 4 millions de Français bénéficient désormais de ce régime. En 2020, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a pris un arrêté rendant plus protecteurs les plafonnements de frais bancaires pour les publics fragiles. En 2022, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré de nouveaux encadrements, notamment pour les Français victimes de fraudes. Parallèlement, Bruno Le Maire s’était engagé, la même année, à instaurer un bouclier tarifaire sur les frais bancaires ; cet engagement a été tenu.

à les encadrer, considérant que la rémunération des services rendus n’est pas un gros mot, mais qu’il faut intervenir pour réglementer quand des excès ou des injustices sont observés. Ce texte prévoit que la gratuité s’appliquera dans trois situations : tout d’abord, pour les comptes dont l’encours est inférieur à 5 000 euros

La facturation de frais bancaires ne sera donc effective et justifiée que dans le cas d’opérations bancaires plus complexes, lorsque les encours sont supérieurs à 5 000 euros. Elle sera assortie d’un plafonnement. Il sera donc possible de ne pas payer de frais bancaires lorsque les encours sont supérieurs à 5 000 euros, si rien ne le justifie. Vous l’aurez compris, nous estimons que ce texte est digne et nécessaire. C’est pourquoi le groupe RDPI soutiendra cette proposition de loi, même s’il préférerait préserver l’équilibre du texte adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. En conclusion, monsieur le ministre, il me semble essentiel que des parlementaires de tous les groupes soient associés aux négociations relatives à la rédaction du décret qui découlera de cette proposition de loi. J’espère qu’il pourra être publié rapidement. Les parlementaires ont pris leurs responsabilités ; désormais, nous comptons sur vous

En effet, en mai 2020, en pleine pandémie, nous avions déjà proposé un dispositif visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires.

Interpellé régulièrement depuis lors, le Gouvernement a lui aussi émis des propositions, mais celles ci sont peu suivies d’actes concrets ou sont insuffisantes face à l’ampleur de l’urgence sociale que nous constatons tous dans le pays. Sur ce même sujet, le texte de notre collègue, la députée socialiste Christine Pires Beaune, que nous étudions aujourd’hui, cible plus particulièrement les frais bancaires en cas de décès et de succession.

Mais là n’est pas l’essentiel. Malgré ces réserves, en fonction bien sûr de la discussion à venir, notre groupe soutiendra la proposition de loi, même modifiée.

à ce texte parce que la poursuite de la discussion parlementaire permettra de nous éclairer sur la position précise du Gouvernement sur ce sujet, et fera émerger, espérons le, un compromis entre les deux chambres du Parlement sur la meilleure rédaction et le meilleur dispositif possible.

C’est un invariant de nos sociétés, peut être même une constante anthropologique. En France, au pays de Descartes, en cette terre de raison, on combine ces deux certitudes : on paie des impôts sur la mort. Je ne parle pas des droits de succession, qui existent dans la plupart des pays ; je parle d’une autre forme de prélèvement obligatoire : les frais bancaires sur les successions. C’est l’association UFC Que Choisir qui a lancé l’alerte en octobre 2021, quelques jours avant la Toussaint, une date choisie.

Au fond, on peut comprendre pourquoi des frais sont prélevés sur ces comptes : les banques doivent procéder à différentes opérations liées à leur clôture, ce qui peut mobiliser des ressources et donc coûter de l’argent. On comprend moins bien, en revanche, pourquoi ces opérations seraient à ce point plus coûteuses en France qu’ailleurs. On peut aussi se demander, et ne pas comprendre, pourquoi une banque ferait payer son décès à un client. décès à un client. On nous parle souvent des incidences comportementales des frais bancaires : par exemple, prélever des agios inciterait les clients à ne pas avoir un compte à découvert. Mais dans le cas d’un défunt, on voit mal ce qui est attendu de lui… La question de l’interdiction pure et simple de ces frais se pose donc. Elle a d’ailleurs été posée ! Mais c’est ignorer en partie la réalité : interdire purement et simplement aux banques de prélever des frais sur les comptes des défunts revient en fait à contraindre les banques à reporter les coûts liés à la succession sur les comptes d’autres clients. C’est pourquoi il nous paraît plus juste d’encadrer ces frais de façon mesurée et raisonnable. En répartissant de façon plus équitable les coûts entre les clients, on évite de matraquer les petits patrimoines, on empêche le prélèvement de frais trop élevés sur des sommes modestes 300 euros de frais bancaires pour moins de 5 000 euros d’encours, il faut le dire, c’est une forme de taxe sur le deuil. C’est ce mécanisme que le Sénat avait adopté, il y a un peu plus d’un an, voté l’excellente proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants. Ce texte, déposé par notre rapporteur général, Jean François Husson, et par son prédécesseur, Albéric de Montgolfier, n’a malheureusement pas prospéré.

de loi. Nous étions donc prêts à légiférer sur la question. J’en profite pour saluer la détermination du Gouvernement qui, après avoir temporisé, a choisi d’inscrire ce texte d’initiative parlementaire à l’ordre du jour, dans une semaine qui lui est réservée. de loi que je viens d’évoquer, avait indiqué qu’il souhaitait éviter une solution législative à un problème qui, somme toute, aurait pu être directement réglé par les banques. Cette solution n’est pas advenue et vous en avez, monsieur le ministre, tiré toutes les conséquences. Notre groupe se réjouit que la loi évolue bientôt en ce sens. La parole

d’expérience – des gens malintentionnés ou oublieux ont tendance à réclamer une deuxième fois des frais d’obsèques qui, pourtant, ont déjà été payés. Je vous assure que c’est un sujet

Écologiste – Solidarité et Territoires salue la proposition de loi de notre collègue députée Christine Pires Beaune, que nous examinons aujourd’hui et qui permet d’engager – enfin ! – un encadrement des frais pratiqués par les établissements bancaires sur les successions. les successions. Depuis 2021, l’UFC Que Choisir a lancé la publication annuelle d’études pour documenter le phénomène. Pour les successions de 20 000 euros, il s’avère que ces frais s’échelonnent entre 80 euros et 527 euros en fonction des établissements bancaires et ils ont connu une croissance de 50 % depuis 2012 et, surtout, de 25 % depuis 2021, soit des niveaux sensiblement supérieurs à l’inflation, alors même qu’il est communément admis que les tarifs imposés sont totalement décorrélés des frais réels engagés par les établissements bancaires.

sont librement déterminées par les établissements bancaires et que l’absence de règles autorise les banques à fixer des prélèvements sur les successions variant du simple au quadruple et à des niveaux deux à trois fois supérieurs à ceux qu’on observe dans le reste de l’Union européenne. proposition de loi en première lecture au Sénat est donc une bonne nouvelle et son adoption dans quelques minutes une première pierre utile dans la régulation des frais bancaires sur succession et même, j’ose le dire, dans la régulation des frais appliqués par les banques.

disproportionnés qui continuent d’enrichir une poignée d’actionnaires au détriment des plus précaires, qui vivent, ou plutôt survivent, à découvert et doivent trop souvent s’acquitter de frais prohibitifs – cela concerne 18 % de la population J’en termine sur le texte de la commission. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires était davantage favorable à la proposition de loi telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais il soutiendra le texte modifié par le Sénat aujourd’hui. Nous émettons une réserve sur le fait d’introduire dès maintenant une limite de 1 % de prélèvement maximal pour la clôture du compte lors des successions dites complexes. De la même manière que la commission a jugé inopportun le seuil de 5 000 euros pour les successions modestes, la fixation dans la loi du seuil de 1 % pour le niveau maximal de frais applicables sur une clôture de compte présente, selon nous, un risque : ce seuil, assez élevé, pourrait conduire les banques à appliquer, à la suite de l’adoption de ce texte, des tarifs rehaussés par rapport aux niveaux actuels. Comme le souligne notre collègue Rémi Féraud dans son amendement n° 1 – un amendement que nous soutiendrons –, la voie réglementaire est plus adéquate pour distinguer plus finement les différents cas de figure et permet davantage de souplesse

Comme sur un grand nombre de sujets, l’exécutif promet, mais n’agit pas. En janvier 2022, Bruno Le Maire promettait une solution rapide. En septembre 2022, il promettait de nouveau une solution – ce devait être pour l’automne. En janvier 2023, la Gouvernement promettait un accord de de place sous un mois. Finalement, rien n’a émergé ! Cette proposition de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale est donc la bienvenue. Elle s’inspire très largement d’une proposition de loi portée par la majorité sénatoriale en 2022, notamment par notre rapporteur Hervé Maurey, dont je tiens à saluer l’opiniâtreté. Elle a été adoptée à l’unanimité par les députés et a été utilement précisée et complétée par notre commission des finances. Elle va permettre de supprimer les frais bancaires prélevés sur les successions soit lorsque le défunt était mineur, soit lorsque la succession représente un montant faible, montant fixé par voie réglementaire, soit lorsque la succession est suffisamment simple pour faire l’objet d’une procédure de clôture de compte simplifiée. Dans les autres cas, des frais pourront être prélevés. Ils seront fixés par décret et ne pourront pas excéder 1 % du montant total figurant sur les comptes du défunt. Sur ce point, je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, pour savoir précisément de quels frais il s’agit. l’article L. 312–1–7 du code monétaire et financier prévoit que « la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite ». Dans sa proposition de loi de 2022, notre rapporteur précisait que cet article s’appliquait à la clôture d’un compte du vivant du client. En effet, cet article se rapporte à une sous section du code monétaire et financier intitulée « Relations des établissements de crédit avec le client » et ne concernerait donc pas l’héritier, qui n’est pas le client de la banque. Mais, à l’Assemblée nationale, votre collègue du Gouvernement, Olivia Grégoire, a indiqué : « L’encadrement tarifaire recherché concerne les opérations bancaires liées à la succession […] qui précèdent nécessairement l’action de clôture des comptes du défunt, dont la gratuité est garantie […] dans le code monétaire et financier. Selon la ministre, la clôture des comptes du défunt est donc gratuite. Seules les opérations préalables seraient concernées. Elle a cité notamment le blocage des comptes, la liquidation des produits d’épargne ou encore la vérification des pièces portées par le successible. Il me semble donc qu’il y a là une légère différence d’interprétation entre le Gouvernement et notre rapporteur. Monsieur le ministre, merci de bien vouloir éclaircir ce point. Pour conclure, nous estimons que le point d’équilibre auquel nous sommes parvenus est satisfaisant. D’un côté, prélever des frais, parfois de l’ordre de plusieurs centaines d’euros, sur le compte d’un défunt quand celui ci ne va ne va transmettre que 1 000 ou 2 000 euros ou lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant apparaît quelque peu déplacé. Même si une succession entraîne un certain nombre d’opérations pour l’établissement bancaire, il nous semble que celui ci peut accompagner gratuitement les héritiers les plus défavorisés, des parents endeuillés, ou dans les cas les plus simples. D’un autre côté, dans les cas plus complexes, il est vrai que les démarches à entreprendre par les banques peuvent être assez lourdes, avec des services parfois non automatisables, et peuvent durer plusieurs mois. Cela entraîne nécessairement un coût en termes de temps passé sur le dossier. Il est donc justifié que des frais soient appliqués, dans une limite définie. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi telle qu’améliorée par notre Haute Assemblée.

par cette proposition de loi, notamment le fait que cela s’applique bien aux héritiers. C’est tout l’intérêt de cette proposition de loi et je crois que cela clarifie le débat juridique qui a existé – vous avez raison de le rappeler. Ce texte permet de définir le champ concerné. L’avis est

qui prévoit la gratuité pour les enfants mineurs décédés. Vous savez, j’ai été maire d’une commune rurale pendant une quarantaine d’années et, dans un petit village, on est au cœur de la douleur. J’ai vu des parents perdre des enfants, j’ai vu des parents perdre des adolescents, j’ai vu des parents perdre des garçons ou des filles de 22 ans, de 25 ans… Je peux vous assurer

Actuellement, malgré les dispositions du code monétaire et financier, il y a deux choix possibles dans le traitement du versement des fonds issus de successions comportant de multiples héritiers, et ce quel que soit le montant de ces fonds.

les répartir auprès des autres héritiers. En cas de mésentente entre héritiers, l’établissement bancaire renvoie alors la répartition des fonds vers un notaire, cette saisine pouvant générer des frais.

dans le cas de successions qui ne sont pas réglées. Cela déstabiliserait complètement la manière dont les successions sont réglées dans notre pays. Nous ne pouvons pas demander aux établissements bancaires d’endosser une telle responsabilité.

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

en la matière, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). Ce texte a été appliqué pendant plusieurs années avant de faire l’objet d’une évaluation

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi dont l’ultime étape de l’examen parlementaire nous réunit ce soir marque une nouvelle avancée importante pour renforcer un volet majeur de notre arsenal de lutte contre la criminalité organisée : la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait abouti à un texte dont les dispositions justes et efficaces font largement consensus. À cet égard, je tiens d’emblée à souligner l’engagement de la rapporteure, Mme Muriel Jourda, que je salue. Ce consensus est, je le crois, le reflet de celui qui traverse la société sur la nécessité d’adopter des mesures fortes afin de toujours mieux lutter contre le crime organisé, sur tous les fronts.

pour les règlements de comptes, la création d’un véritable statut de repenti, ou encore celle d’un crime d’association de malfaiteurs, puni de vingt ans de réclusion. Ce n’est bien sûr pas l’objet du texte qui nous occupe ce soir, mais je tenais à le mentionner pour replacer cette proposition de loi dans le cadre d’une action globale, forte et volontariste, à laquelle elle contribue de manière tout à fait substantielle. Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner et ainsi donner corps à l’adage selon lequel le crime ne paie pas a a toujours constitué un axe majeur de la politique pénale du Gouvernement. Notre arsenal législatif a évolué en ce sens pour favoriser l’engagement des enquêteurs et des magistrats, qui saisissent et confisquent toujours plus. Je salue leur action qu’illustrent les chiffres records d’une politique pénale parfaitement intégrée : les saisies réalisées en 2023 s’élèvent à 1,44 milliard d’euros et ont été multipliées par dix depuis 2011, tandis que le montant des confiscations prononcées a atteint le chiffre inégalé de 175,5 millions d’euros, soit une augmentation de 105 % en trois ans.

En somme, le dispositif de saisie et de confiscation des avoirs criminels a régulièrement été amélioré, car frapper les délinquants au portefeuille est triplement gagnant. Oui ! C’est une arme extrêmement puissante de répression cela renforce l’indemnisation des victimes ; et cela envoie un message de fermeté particulièrement dissuasif. Le texte que vous allez, je l’espère, adopter définitivement tout à l’heure donnera un nouvel élan à cette dynamique vertueuse, en nous dotant de moyens à la hauteur de l’enjeu et de nos ambitions. Avant de revenir rapidement sur les principales dispositions du texte, je tiens à saluer le travail qui a été mené en commission mixte paritaire pour tenir compte des nombreux enrichissements venant tant de l’Assemblée nationale que du Sénat, comme des exigences constitutionnelles et des difficultés pratiques auxquelles les magistrats sont confrontés. En effet, pour donner leur plein effet aux procédures de confiscation, il convient avant tout de les rendre suffisamment simples et suffisamment pratiques pour que les magistrats puissent efficacement s’en emparer.

Concrètement, cela veut dire que les biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction seront systématiquement saisis. Cela constitue un tournant important dans la pratique judiciaire, qui renverse la logique qui prévalait jusque là. sauf décision motivée, la juridiction doit confisquer, afin de s’assurer que le crime ne paie plus, et que bien mal acquis ne profite jamais. Une autre avancée mérite d’être soulignée. La proposition de loi a élargi l’affectation avant jugement des biens saisis au profit des services judiciaires, de l’administration pénitentiaire et des établissements publics sous tutelle du ministère de la justice, parmi lesquels l’Agrasc. Je tiens également à revenir sur un apport important du Sénat, qui comble une lacune qui a été révélée par la pratique, à savoir l’absence d’acteur judiciaire désigné pour statuer sur les biens une fois la juridiction de jugement saisie.

que soit désigné un magistrat compétent, à savoir le président du tribunal judiciaire ou un juge désigné par lui, pour statuer sur le sort des biens saisis une fois que la juridiction de jugement a été saisie.

Enfin, la confiscation d’un immeuble constituera désormais un titre d’expulsion à l’encontre du propriétaire condamné et de sa famille. Seul le locataire de bonne foi sera protégé. Les proches du délinquant ou du criminel ne pourront plus profiter de l’immeuble saisi et en seront chassés.

Il incarne cette justice vertueuse qui rassemble, qui protège et qui nous oblige. Je tiens une fois encore à saluer les rapporteurs, le député Jean Luc Warsmann et la sénatrice Muriel que l’ensemble des sénateurs et des députés de tous bords qui se sont investis sur ce texte. L’engagement du Gouvernement pour lutter contre la délinquance et la criminalité reste total, et cette proposition de loi y contribue résolument en faisant un pas supplémentaire dans la bonne direction. C’est pourquoi je vous invite à l’adopter largement. je vous remercie

Cette loi a offert de larges possibilités opérationnelles et a permis de prononcer des sanctions patrimoniales significatives. Puis les différentes évolutions législatives

Je pense, en particulier, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Je tiens à souligner et à saluer le travail de cette agence au cours de sa première décennie d’exercice, puisque le nombre de saisies enregistrées a constamment augmenté, année après année. Pourtant, dans leur rapport de 2019, les députés Laurent Saint Martin et Jean Luc Warsmann ont souligné le paradoxe qui entoure les procédures de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Selon leurs conclusions, nous sommes dotés d’un cadre législatif élaboré, mais dont les mécanismes demeurent très insuffisamment utilisés. Ils déploraient également le fait que l’utilisation des techniques d’identification des avoirs criminels et le recours aux saisies étaient trop concentrés sur les affaires économiques et financières et les affaires

Cette proposition de loi nous invite donc à aller plus loin. Au nom de mon groupe, je soutiens les différents dispositifs qu’elle comporte. Je pense naturellement aux dispositions initialement proposées, par exemple à l’article 1, modifie la procédure de contestation des décisions de saisie de biens meubles prises avant jugement, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Je pense aussi à l’article 2, qui simplifie l’indemnisation des victimes dans la gestion des biens confisqués. L’article 3 comprend également de très bonnes mesures, telles que la confiscation systématique et de plein droit des biens lorsqu’ils « ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou Je me réjouis que notre assemblée ait su doter le texte de nombreux apports. Par exemple, l’article 1 , qui comble une lacune juridique dans la gestion des biens saisis entre la fin de l’enquête ou de l’instruction et la tenue de l’audience de jugement, de même pour l’article 2 A, que le Sénat a adopté en séance publique et qui prévoit l’extension du champ de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à une série de nouvelles infractions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer revêt une importance cruciale. Il vise à améliorer l’efficacité l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, et contribue ainsi à donner encore plus corps à l’adage selon lequel nul ne doit tirer profit de son crime. Ces dispositifs constituent des leviers puissants lutter contre la criminalité organisée, dont il est avéré que les acteurs craignent souvent plus pour leur portefeuille que pour leur liberté. C’est donc à leur portefeuille qu’il convient de les frapper, et de les frapper fort, en réaffirmant avec conviction que le crime ne paie pas. Le respect de ce principe est d’autant plus important qu’il conditionne l’efficacité et la crédibilité de la réponse pénale. À cet égard, les mécanismes actuels de saisie et de confiscation, qui reposent largement sur les dispositions de la loi Warsmann du 9 juillet 2010, ont largement prouvé leur redoutable efficacité. Je rappelle que, depuis la création de l’Agrasc, le montant des saisies n’a cessé d’augmenter : de 109 millions d’euros en 2011, il est passé à 1,44 milliard d’euros d’euros en 2023, tandis que le montant des avoirs confisqués s’élevait à 175 millions d’euros. Si ces chiffres sont encourageants, il faut reconnaître que subsistent d’importantes marges de progression. Ainsi, seuls 30 % des biens saisis finissent par être effectivement confisqués. Il faut donc aller plus loin.

qui a présidé à l’examen de ce texte, tout au long de la navette parlementaire, et qui a permis d’aboutir, en commission mixte paritaire, à un texte consensuel auquel notre chambre a largement contribué.

complémentaire de confiscation générale du patrimoine ; l’extension de la possibilité de remise à l’Agrasc des biens meubles confisqués. Le travail pragmatique mené par les deux chambres, en bonne intelligence avec le Gouvernement, nous a permis d’aboutir à un texte équilibré et efficace, dont je ne doute pas une seconde qu’il permettra aux mécanismes de saisie et de confiscation d’atteindre leur plein potentiel. C’est en conséquence avec beaucoup d’enthousiasme que les élus du groupe RDPI voteront en faveur de cette

même si nous regrettons que nos amendements inspirés par Transparency International et Crim’Halt n’aient pas été repris en première lecture.

permettre la fermeture administrative des commerces de façade qui pullulent dans certains quartiers, au vu et au su de tous, et qui constituent de véritables lessiveuses.

nous nous réjouissons du caractère conclusif de la CMP réunie le 30 avril dernier. Le fruit de ce travail mené en commun nous semble aussi pertinent qu’indispensable dans la lutte contre le crime. Ce texte de loi renforcera incontestablement notre arsenal législatif. Grâce à lui, nous pourrons mieux appréhender le patrimoine des délinquants et des criminels.

L’autre apport majeur du texte, que nous devons à notre rapporteur, chère Muriel Jourda, consiste dans la possibilité de gérer les biens saisis à l’issue de l’enquête ou de l’instruction avant que le tribunal n’ait statué sur le sort de ces derniers.

passera également par la désignation, dans la loi, d’un acteur judiciaire qui statuera sur les biens une fois la juridiction de jugement saisie. Ainsi, le président du tribunal judiciaire, ou un juge délégué par lui, aura compétence pour statuer sur les requêtes relatives à l’exécution de la saisie des biens. En outre, le compromis trouvé en CMP au sujet de l’article 3 nous paraît très pertinent. Il facilitera – nous l’espérons – l’expulsion des personnes occupant de mauvaise foi un logement confisqué par la justice. pas non plus la place des victimes : nous nous félicitons de l’allongement du délai leur permettant de demander l’obtention des biens confisqués. Le délai de deux mois était bien trop court ; un délai de six mois facilitera la réponse à leurs requêtes.

rendre hommage à l’action déterminante des policiers, des gendarmes, des douaniers, des magistrats et bien sûr des équipes de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Non, le crime ne doit plus enrichir impunément ! Nous saluons la rigueur et la précision du travail mené sur ce sujet à la fois technique et essentiel par notre rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels sont aujourd’hui des outils essentiels pour préserver l’ordre public, la sécurité et la justice.

un moyen de dissuader ceux qui seraient prêts à s’engager dans des activités illégales et de réparer les dommages subis par les victimes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous présentions hier le rapport de la commission d’enquête sur le narcotrafic, qui inclut un certain nombre de préconisations visant à améliorer l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation. On constate que, plus que jamais, nous avons besoin d’une réflexion législative allant au delà du tout prison. Je regrette d’ailleurs que nous n’ayons pu attendre les conclusions de cette commission d’enquête pour légiférer en la matière. Je salue la qualité des travaux menés par son président, Jérôme Durain, et par son rapporteur, Étienne Blanc. Leur rapport contient, entre autres, trois préconisations directement instaurer une procédure de gel administratif et de saisie conservatoire des biens des narcotrafiquants ; autoriser la confiscation sans condamnation pénale ; faciliter la saisie des fonds de commerce. Quels que soient les méfaits commis – délinquance financière, narcotrafic, etc. –, les délinquants détestent être frappés au portefeuille.

au 30 septembre 2023, 57,6 % l’avaient été dans le cadre de dossiers comprenant au moins une infraction à la législation sur les stupéfiants ». De même, ce travail met en lumière l’importance de la formation des agents à tous les niveaux [l]es juridictions qui bénéficient du soutien d’assistants spécialisés ou de juristes assistants assurant la formalisation et le suivi des décisions de saisies pénales sont plus dynamiques en matière de saisies et de confiscations.

devant la chambre de l’instruction. La contestation des décisions de saisie représente actuellement 40 % du contentieux dans certaines chambres d’instruction. L’article 1 allège le contentieux en permettant de procéder aux contestations auprès du premier président de la cour d’appel. Dans cette même veine, nous accueillons favorablement les précisions apportées à l’article 3 afin de simplifier les procédures, qui enrayent parfois la machine, sans pour autant obérer les droits du justiciable.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Il faut taper les délinquants au portefeuille. » Dès 1982, l’Italie créa un dispositif juridique de saisie et de confiscation des avoirs criminels, par la loi dite Pio La Torre, du nom du célèbre député communiste sicilien. qui paya de sa vie sa lutte contre la mafia, laissa en héritage le premier dispositif de confiscation obligatoire des biens criminels. En France,

Puis, en 2021, deux textes sont venus compléter cet arsenal, en facilitant la saisie et l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués et en instituant un mécanisme de restitution des biens mal acquis l’aide au développement.

En effet, malgré la progression fulgurante des saisies et des confiscations, nous demeurons loin des résultats atteints par l’Italie, qui a confisqué plus de 11 milliards d’euros de biens à la mafia au cours des vingt dernières années et qui a généralisé l’usage social Grâce à cette proposition de loi, le volet répressif et dissuasif du mécanisme de saisie et de confiscation des avoirs criminels est renforcé. Les saisies seront désormais plus rapides, plus efficaces,

En outre, la confiscation obligatoire est étendue non seulement aux biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, mais également aux biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

l’exemple de l’Italie est inspirant : pour la seule année 2019, 947 biens criminels ont été mis au service de l’économie sociale et solidaire. Ils ont à 505 associations ou organismes d’HLM, à 26 fondations, à 27 écoles, à 16 associations sportives et à 5 organismes de formation professionnelle. Mes chers collègues, mettre les biens criminels au service de l’intérêt général, c’est rendre aux citoyens les fruits du crime organisé et démontrer que les systèmes mafieux ne l’emportent pas sur la défense du bien commun. C’est ainsi que nous réparerons les dommages commis par le crime dans nos territoires. Nous saluons pleinement cette proposition de loi, car nous sommes bien de ceux qui pensent que ce qui fait l’efficacité de la peine, ce qui la rend dissuasive, ce n’est pas sa sévérité, mais sa certitude. je vous remercie

monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons une nouvelle fois devant le Sénat pour l’examen d’un texte d’apparence très technique, mais dont les effets seront, dès sa promulgation, très concrets pour bon nombre de nos concitoyens. Son adoption est essentielle pour assurer la pérennité de plusieurs évolutions récentes de notre droit dans les collectivités du Pacifique. En effet, le 19 avril dernier, le Gouvernement a étendu et adapté par ordonnance plusieurs mesures du code de la santé publique déjà en vigueur dans l’Hexagone et dans les départements et régions d’outre mer, afin qu’elles puissent s’appliquer en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, en tenant compte, bien sûr, de l’organisation particulière de ces territoires. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 74 1 de la Constitution, qui prévoit une habilitation permanente du Gouvernement pour étendre à l’outre mer les dispositions législatives déjà existantes et qui relèvent de la compétence de l’État. La contrepartie évidente de cette habilitation permanente est que les ordonnances prises sur ce fondement doivent être nécessairement ratifiées par le Parlement, ce qui implique un projet de loi spécifique et justifie ma présence devant vous cet après midi. En effet, En effet, faute d’une ratification expresse par les parlementaires dans un délai de dix huit mois, l’ordonnance deviendrait caduque. Dans la mesure où ses dispositions ont pris effet dès leur publication, le présent projet de loi a pour objet non pas de modifier le droit pour l’avenir, mais bien d’assurer la pérennité des modifications apportées au code de la santé publique. Concrètement, une absence de ratification entraînerait un retour au droit antérieur pour nos concitoyens du Pacifique sur les thématiques visées par l’ordonnance. Une telle régression concernerait des sujets d’importance ; elle serait bien sûr regrettable. Le premier objet de cette ordonnance est en effet de rattraper un certain retard en matière d’applicabilité des lois de bioéthique en rendant applicables dans les trois collectivités du Pacifique les récentes dispositions du code de la santé publique se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine dispositions permettent de préciser les conditions dans lesquelles peuvent être menées ces recherches et de garantir la sécurité et la bonne information du participant. En adaptant à ces territoires le droit applicable en la matière, tel qu’il est issu des dernières évolutions législatives à l’échelon national et européen, le Gouvernement pose un cadre sécurisant qui va permettre le développement de telles recherches dans les collectivités du Pacifique. De plus, l’ordonnance étend et adapte diverses dispositions législatives relatives à la santé, dans le respect des partages de compétences entre l’État et chacune de ces collectivités. C’est notamment le cas de certaines dispositions de la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement. Je pense en particulier à l’allongement des délais de recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) de douze à quatorze semaines et à la suppression du délai minimal de réflexion à l’issue d’un entretien psychosocial, étant entendu que vous avez voté en Congrès, il y a quelques mois à peine, l’inscription dans notre Constitution de la liberté de recourir à l’IVG. L’unification des règles de recours en la matière vise ainsi à améliorer et à sécuriser l’effectivité du droit des femmes à pleinement disposer de leur corps dans tous les territoires de la République. aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, qui étendent les compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles de la Polynésie française, l’ordonnance y étend les dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé relatives à la protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures. Là encore, l’objectif du Gouvernement, par cette ordonnance, est de sécuriser des mesures législatives importantes pour l’accès à la santé et à la prévention, de sorte que l’ensemble de nos concitoyens Enfin, dans le même souci de garantir une application uniforme du droit en matière de santé sur tout le territoire, un amendement déposé par le Gouvernement a été adopté par l’Assemblée nationale pour étendre à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française l’article L. 1243 6 du code de la santé publique, qui définit les lieux dans lesquels peuvent être réalisées les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi vous est soumis après un nouvel examen attentif par votre commission des affaires sociales. affaires sociales. Je suis certain que notre objectif trouvera un écho favorable dans votre chambre, car, je le répète, il s’agit d’assurer la pérennité de mesures utiles et importantes concernant notamment les recherches impliquant la personne humaine ou les délais de recours

pour examiner en deuxième lecture le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé. Je le rappelle, le premier objet de cette ordonnance était de rendre applicables dans ces territoires certains volets des dernières lois de bioéthique en matière de recherche, en particulier les dispositions du code de la santé publique se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine.

article unique se bornait à prévoir la ratification nécessaire de l’ordonnance précitée, prise sur le fondement de l’article 74 1 de la Constitution.

Le Sénat avait ensuite adopté ce texte en séance publique sans modification. En première lecture, l’Assemblée nationale a quant à elle adopté conforme l’article unique, devenu article 1, procédant à la ratification de l’ordonnance du 19 avril 2023.

Ce nouvel article vise notamment à répondre aux demandes d’adaptations complémentaires du code ou de corrections de malfaçons législatives formulées par la Nouvelle Calédonie et par la Polynésie française. Celles ci concernent principalement la déclinaison territoriale de dispositions relatives à l’organisation des soins, à l’assistance médicale à la procréation (AMP) ou aux recherches impliquant la personne humaine. Ajouté sur l’initiative de Mme Reid Arbelot, l’article 3 dispose : « Dans un délai

L’Assemblée nationale ayant adopté conforme l’article 1, nous devons nous prononcer aujourd’hui sur les deux seuls articles nouveaux, qui restent en discussion. Vous le savez, j’avais regretté que les adaptations complémentaires demandées par les territoires n’aient pu être prises en compte au stade de la première lecture au Sénat. J’avais sollicité le ministère de la santé, en amont de l’examen du texte en commission,

J’avais également interpellé, en séance publique, la ministre Fadila Khattabi sur ce sujet. Celle ci avait alors renvoyé ces modifications à un examen ultérieur, invoquant des délais trop tardifs. Les modifications finalement intervenues à l’Assemblée nationale quelques semaines plus tard ne font que démontrer, une fois de plus, la méthode discutable que le Gouvernement a adoptée à l’endroit du Parlement.

sans être prêt, le Gouvernement nous contraint aujourd’hui à nous résoudre à une deuxième lecture. Vous en conviendrez, monsieur le ministre : une lecture dans chacune des chambres aurait normalement permis de répondre convenablement aux besoins. Ces réserves de méthode mises à part, la commission des affaires sociales a approuvé les modifications ainsi apportées au code de la santé publique. Il s’agit de clarifier les adaptations applicables et de tirer les conséquences, dans l’application ou non de certaines dispositions, de la compétence dévolue en matière de santé à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française. Je suis consciente que ces aménagements ne répondent pas à l’ensemble des demandes des territoires. Cependant, ils me semblent correspondre à une interprétation efficace du partage de compétences entre l’État et le « pays L’article 2 participe ainsi de la mise à jour attendue du droit de la santé et de la recherche. J’en viens à l’article 3. Vous le savez, la commission des affaires sociales est par principe défavorable aux demandes de rapport.

Surtout, la commission n’a pu que se résigner à faire le constat d’une demande de rapport mal définie. Son champ territorial ne se limite ainsi pas expressément aux seules collectivités du Pacifique, alors qu’aucune disposition du présent texte ne vise le droit commun et qu’il ne relève donc pas de ce projet de loi de prévoir l’évaluation d’une politique nationale. même du texte, la commission regrette sa focalisation sur un aspect financier, qui n’est qu’un prisme restreint de lecture des difficultés opérationnelles de mise en œuvre de l’extension de l’allongement du délai de recours à l’IVG. Tel n’est sans doute pas, d’ailleurs, le problème visé. Les questions soulevées sont en réalité plurielles, au delà du seul coût budgétaire : adaptations juridiques, compétences des professionnels, règles de prise en charge, enjeux de formation, structures et professionnels de santé disponibles.

la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française les récentes dispositions du code de la santé publique se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine, à l’allongement du délai de recours à l’interruption volontaire de grossesse ou encore à l’organisation et à la réalisation des soins. pour les dispositions portant extension des compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles aux îles Wallis et Futuna, mais aussi aux mesures relatives à la protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures en Polynésie française. Bien que ces avancées législatives soient le fruit de combats politiques menés par la majorité présidentielle depuis 2017, notre rôle, aujourd’hui, est purement légistique. Les débats politiques autour de ces questions de fond n’ont pas lieu d’être, car ils ont déjà été menés.

Ce texte permet à toutes les Françaises et à tous les Français, où qu’ils se trouvent sur le territoire national, d’avoir les mêmes droits dans le domaine de la santé. Il donne accès aux habitants des collectivités du Pacifique à des traitements innovants

Elles ont été satisfaisantes : elles ont permis de préciser la portée de la ratification et d’enrichir de façon bienvenue le travail parlementaire. Il convient désormais d’adopter conforme le texte ainsi modifié.

n° 2023 285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé

l’application des nouvelles dispositions relatives à la bioéthique, mais aussi des règlements européens portant sur les essais cliniques de médicaments, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic . L’on L’on ne peut que regretter que les territoires français du Pacifique aient dû attendre plus de dix ans pour disposer d’un cadre juridique adapté en matière de bioéthique – les lois de bioéthiques ont été votées en 2012

; suppression du délai minimum de réflexion de deux jours pour confirmer un avortement ; possibilité de recourir à la téléconsultation pour l’avortement ; autorisation accordée aux sages femmes de réaliser des IVG par voie instrumentale dans les établissements de santé ; élargissement des compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles chez les partenaires des femmes. Toutes ces dispositions ont pour but d’améliorer le système de santé en favorisant la confiance et la simplification des procédures.

et compassionnel à certains traitements, évolutions issues des lois de financement de la sécurité sociale pour 2021 et pour 2022. Des patients en impasse thérapeutique peuvent ainsi bénéficier à titre exceptionnel et temporaire de certains médicaments non autorisés dans une indication thérapeutique précise. Des médicaments sans autorisation de mise sur le marché peuvent être utilisés pour traiter des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié, que le patient ne peut être inclus dans un essai clinique et que la mise en œuvre du traitement ne peut être différée. Monsieur le ministre, disposez vous de données nous permettant de mesurer la qualité de la prise en charge des patients ultramarins qui Autre disposition positive contenue dans l’ordonnance du 19 avril 2023 : l’application à la Polynésie française de la possibilité offerte à un plus grand nombre de professionnels de santé de déroger à l’obligation de recueillir le consentement de l’autorité parentale dans des situations où des actions de prévention, de dépistage ou de traitement

de ratifier l’ordonnance du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé.

Elles comportent notamment des mesures de rattrapage en matière de recherche sur la personne humaine en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. En tant que sénateur ultramarin, je souhaite saluer ces évolutions, car, en l’état car, en l’état actuel du droit, la Polynésie française ne pouvait contribuer à ces RIPH, tandis qu’en ce domaine les possibilités de la Nouvelle Calédonie étaient limitées.

par les gouvernements de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie. Faute de temps, ce travail n’avait pu être entrepris avant la première lecture au Sénat : c’est désormais chose faite. qui permet de parfaire le dispositif de l’ordonnance et de corriger autant que possible les imperfections du code de la santé publique tel qu’il s’applique dans nos territoires du Pacifique.

ainsi ratifiées permettront notamment de confier aux autorités locales la définition de l’équipe de soins intervenant auprès d’un patient. Elles conféreront aux autorités du pays le pouvoir de décider de l’organisation des professionnels ou ou organismes concourant à la prévention ou aux soins et produisant des documents comportant des données de santé à caractère personnel. Elles permettront à la Polynésie française de bénéficier des règles applicables à l’État en matière de promotion des recherches

peuvent être réalisées les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire. Les dispositions que nous étudions sont techniques, mais elles permettront d’adapter et de moduler celles que nous avions entérinées en adoptant l’article 1, qui permettaient déjà de rattraper un retard accumulé depuis plus de dix ans en matière de santé et de recherche dans les outre mer.

le projet de loi de ratification qui nous est soumis va dans le bon sens. L’adoption de l’article 1, le 14 mars dernier, permet de rendre applicables aux îles Wallis et Futuna,

portant sur les essais cliniques de médicaments, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic , dans le respect de leur statut européen de pays et territoires d’outre mer. Cette ordonnance a aussi vocation à acter des avancées particulières pour les îles Wallis et Futuna, à commencer par les dispositions visant à renforcer le droit à l’avortement.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la Polynésie française, cette ordonnance y apporte, outre les mêmes avancées relatives à l’IVG, une meilleure protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures, ou encore de nouvelles garanties en matière de données des patients. Comme l’avait déjà souligné ma collègue Lana Tetuanui le 14 mars dernier, nous approuvons ces avancées pour la protection et la liberté des femmes, mais encore faut il que les moyens suivent. Or nous connaissons parfaitement les difficultés que rencontrent les structures médicales en Polynésie, comme d’ailleurs Nous devons aujourd’hui nous prononcer sur deux nouveaux articles ajoutés par nos collègues députés. Je partage à ce sujet le sentiment exposé il y a quelques instants par notre rapporteure.

Ces demandes concernent des adaptations ou des corrections de malfaçons législatives : il s’agit de rendre la plus juste possible la déclinaison territoriale des dispositions relatives à l’organisation des soins, à l’assistance médicale à la procréation ou aux recherches impliquant la personne humaine. Même si, sur la

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, il est impossible pour notre groupe de commencer cette intervention sans exprimer notre plus profonde inquiétude face à la situation de la Nouvelle Calédonie, ce que nous n’avons pas pu faire au Gouvernement. Nous condamnons fermement toutes les violences commises et affichons notre soutien plein et entier aux forces de l’ordre et aux habitants de l’archipel. Nous appelons au retour au calme, ainsi qu’au respect des lois de la République.

de la Polynésie française, le projet de loi y assure la mise en œuvre des dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui ont trait à la protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures. Ainsi, nous sécurisons et renforçons le droit des femmes d’outre mer à disposer de leur corps. Enfin, conformément à la répartition des compétences dans ce territoire, cette ordonnance étend à Wallis et Futuna les seules dispositions relatives à l’extension des compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles. Sur la forme, nous regrettons, tout comme notre rapporteure, que ce texte ait été inscrit à l’ordre du jour avant que ne soit achevé le travail de concertation avec les territoires, ce ce qui nous contraint aujourd’hui à une deuxième lecture quand une seule aurait pu suffire. Depuis le premier examen de ce projet de loi par la Haute Assemblée, de nombreuses modifications sont intervenues. Il s’agit surtout d’adaptations du code de la santé publique concernant la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française ou de corrections de dispositions qui ne tenaient pas compte des nécessités d’adaptation à ces territoires. Les modifications apportées à la version que nous avons votée au mois de mars en disent long sur la complexité du droit des outre mer ; elles témoignent également de la nécessité de faire preuve de la plus grande rigueur dans l’application de notre corpus législatif dans ces

s’il faut étendre ou non les règles applicables dans l’Hexagone à ces territoires, mais de déterminer si celles ci pourront effectivement y être appliquées, compte tenu des moyens humains et matériels disponibles sur place. La situation sanitaire y est parfois alarmante, y compris dans des territoires où l’État est pleinement compétent en matière de santé. C’est pourquoi il nous apparaît impératif de renforcer l’accès aux soins dans toutes les collectivités ultramarines. J’en veux pour preuve l’exemple édifiant de Mayotte, actuellement en proie à une épidémie dramatique de choléra qui s’ajoute aux difficultés chroniques de l’île.

Il y a deux mois, notre assemblée a appelé le Gouvernement à rectifier l’ordonnance en y intégrant les modifications et précisions demandées par les gouvernements de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie, afin de mieux adapter le texte aux spécificités locales,

notamment des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine, des éléments issus de la loi visant à renforcer le droit à l’avortement ainsi que l’extension des compétences des sages femmes en matière de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles. Consultés, les représentants des collectivités ont cependant unanimement regretté les conditions de saisine, qui ne leur ont pas permis de rendre un avis approfondi. Ainsi, seul l’avis du congrès de la Nouvelle Calédonie a été reçu par le Gouvernement la délibération de Wallis et Futuna ne l’a manifestement pas été et l’avis de l’assemblée de la Polynésie française n’a finalement pas pu être formalisé avant la publication de l’ordonnance. Résultat

de ces collectivités. Nous voterons une nouvelle fois le projet de loi ratifiant cette ordonnance, car l’extension de ces dispositions législatives est sans conteste une bonne nouvelle, surtout assortie des modifications nécessaires à une meilleure applicabilité.

seule solution pour ouvrir un véritable dialogue et trouver un accord convenable. Soutenir le choix de l’autonomie du peuple kanak, c’est aussi lui permettre de reprendre en main son propre système de santé et assurer un avenir plus équitable et adapté à ses besoins spécifiques. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l’examen en deuxième lecture de ce projet de loi, nous œuvrons aujourd’hui à ce que le droit s’applique de la même façon à tous les Français et à toutes les Françaises. Il était plus que temps

Nous saluons l’application à ces territoires du Pacifique du secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures, ainsi que la suppression de la notion de détresse pour délivrer la contraception d’urgence. Ces dispositions sont autant de leviers permettant aux femmes de disposer librement de leur corps. Nous saluons aussi les modifications bienvenues apportées par l’Assemblée nationale et issues des demandes émises par la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française, concernant notamment les adaptations complémentaires du code de la santé publique ou la correction de malfaçons législatives.

Pour organiser au mieux ce droit et le rendre effectif, il faut en effet reconnaître son coût pour les collectivités locales qui devront l’assumer et qui connaissent des difficultés budgétaires, comme le savent bien les membres de la chambre haute. nous continuons de dénoncer la méthode utilisée. Je regrette que les conditions complètes du bon examen de ce projet de loi n’aient pas été réunies au mois de mars, quand nous l’avons voté en première lecture, car, alors, le Gouvernement n’avait pas intégré avis transmis par les territoires. La concertation a été bâclée. Si les trois territoires du Pacifique ont été formellement consultés, les délais de saisine ne leur ont pas permis de rendre un avis étayé et complet. Alors que l’ordonnance touche à des sujets de société appelant une consultation élargie de la population, le Gouvernement a saisi l’assemblée de la Polynésie française à la fin du mois de janvier 2023, dans un contexte électoral peu propice à une analyse approfondie. Nous dénonçons toujours le recours aux ordonnances. Ce texte est le reflet de la relégation des outre mer dans l’ordre de la construction de la loi. Trop souvent, la loi s’y résume à des ordonnances d’application prises très tardivement, y compris dans des domaines fondamentaux ; ainsi se trouvent fondées des inégalités entre citoyens. La méthode de l’ordonnance conduit parfois à ce que les droits soient effectifs dans les outre mer des années, voire plus d’une décennie, après leur application dans l’Hexagone. Nous voterons donc pour l’adoption sans modification des dispositions introduites à l’Assemblée nationale, mais nous regrettons qu’il ait fallu attendre si longtemps : nous regrettons que le Gouvernement fasse preuve de beaucoup plus d’empressement et de beaucoup plus de volonté pour imposer par la force le dégel du corps électoral en Nouvelle Calédonie que pour garantir aux femmes et aux hommes des territoires du Pacifique

Monsieur le président, madame la rapporteure, monsieur l’auteur avant d’entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble cet après midi, comment ne pas évoquer la bien triste et tragique actualité de la Nouvelle Calédonie, objet d’un conseil de défense convoqué par le Président de la République ce matin même ? À la suite d’émeutes urbaines, l’état d’urgence a été décrété, alors que l’on déplore la mort de quatre personnes, dont un gendarme, et de nombreux blessés parmi les forces de l’ordre. À qui la faute, demandera t on ? Mais est ce bien le moment de poser cette question alors qu’en Nouvelle Calédonie la paix civile est mise à mal par une explosion dont il faudra, une fois le calme revenu, comprendre les raisons ? Je me contenterai, au nom du groupe du RDSE, d’adresser de sincères condoléances aux proches des victimes et d’appeler à un retour au calme, qui ne pourra se produire que par l’intervention dépassionnée de toutes les forces politiques, locales et nationales. Pour en venir au texte qui nous réunit, l’article 74 1 de la Constitution dispose qu’à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie le Gouvernement peut étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur dans l’Hexagone. C’est dans ce cadre constitutionnel que nous sommes appelés à procéder à la ratification de l’ordonnance du 19 avril 2023 rendant applicables aux trois collectivités françaises du Pacifique les récentes dispositions du code de la santé publique se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine. Cette ordonnance étend également à ces territoires diverses diverses dispositions récentes relatives aux droits des personnes malades, à la santé sexuelle, à l’interruption volontaire de grossesse et à différents produits pharmaceutiques. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette ratification, car il s’agit là d’un simple rattrapage attendu par ces collectivités. Oui à la transposition Oui à la transposition des dernières lois de bioéthique fixant les conditions dans lesquelles des recherches peuvent être engagées et garantissant la sécurité et la bonne information des participants. Oui à l’extension de l’application des règlements européens portant sur les essais cliniques de médicaments, les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic. Oui à la protection par le secret de la prescription de la contraception aux personnes mineures. Oui à l’allongement du délai de recours à l’IVG à quatorze semaines et à la suppression du délai minimum de réflexion à l’issue de l’entretien psychosocial. En revanche, sur la forme, mon groupe l’a indiqué en première lecture et tient à le rappeler, nous déplorons que seul l’avis du congrès de la Nouvelle Calédonie ait été reçu par le Gouvernement dans le délai imparti. Les conditions de saisine des collectivités n’ont pas été satisfaisantes ; elles ne permettent pas toujours de rendre un avis étayé sur le fond ou de mener une analyse juridique fine. de questions techniquement complexes, telles que les recherches impliquant la personne humaine, voilà qui est regrettable. L’Assemblée nationale a introduit deux nouveaux articles qui font l’objet de cette deuxième lecture. Permettez moi de m’interroger, mes chers collègues : ce texte méritait il vraiment une deuxième lecture ? Je n’en suis pas certaine, au regard des urgences que l’actualité nous rappelle.

Sur la demande de rapport, nous partageons également l’avis de la rapporteure : la question n’est pas tant celle du coût de l’allongement du délai de recours à l’IVG que celle des moyens nécessaires pour rendre ce droit effectif partout et pour toutes.

madame la rapporteure, monsieur l’auteur de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie avant tout d’excuser Nicole Belloubet, qui est retenue par ailleurs. Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’examen en deuxième et – je l’espère – dernière lecture de la proposition de loi visant à la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien. Ce texte est très attendu par ces personnels essentiels au fonctionnement de l’éducation nationale que sont les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Je tiens à saluer l’engagement de ces accompagnants ; peut être devrais je dire « de ces accompagnantes », car il s’agit pour une immense majorité de femmes. Ils sont en effet indispensables à notre école et participent en premier lieu à rendre tangible l’école pour tous à laquelle le Gouvernement est extrêmement attaché. L’école dans notre pays doit aujourd’hui faire face à un véritable défi, celui de la prise en compte de l’ensemble des besoins éducatifs particuliers de nos élèves : il s’agit en effet de permettre leur scolarisation à tous, de la maternelle au lycée. L’école, nous le savons, doit être le premier lieu de la solidarité nationale à l’égard des personnes en situation de handicap. Cela implique de faire évoluer, là où c’est nécessaire, les formes de l’enseignement, les relations entre les élèves et les professeurs, l’environnement scolaire et le matériel adapté, en un mot : le quotidien de nos écoles et de nos établissements. C’est là un défi pour l’éducation nationale, mais le Gouvernement y consacre toute son énergie afin d’être au rendez vous. L’institution scolaire doit remplir la mission qui lui est assignée : permettre la réussite et garantir le bien être de tous les élèves dans leur pluralité. Il est toutefois nécessaire également de changer de manière plus profonde le regard que nous portons sur le handicap dans sa diversité. Garantir la continuité de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur toute l’amplitude de la journée d’école, en incluant le temps méridien, est ainsi un pas supplémentaire en faveur de l’inclusion de toutes et de tous dans notre société, en plus d’être une nécessité pour favoriser une scolarité sereine et efficace. Ce défi est d’autant plus grand que le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire est en constante augmentation. L’école et ses professeurs ont donc besoin d’appui.

pour atteindre 86 500 ETP. Je rappelle que le Gouvernement a agi avec force pour que ces personnels soient reconnus comme ils le méritent. Ainsi avons nous revalorisé de manière importante leur salaire, qui a progressé en moyenne de 26 % entre 2021 et 2024, soit 200 euros net de plus par mois. S’il était encore besoin de souligner l’importance de ce métier pour notre école aujourd’hui, je rappellerais également que les AESH sont devenus, en termes d’effectifs, le deuxième métier de l’éducation nationale. Ces progrès étaient donc attendus et nécessaires ; nous en sommes fiers. La proposition de loi qui vous est soumise aujourd’hui s’inscrit pleinement dans cette dynamique : elle prévoit la prise en charge à 100 % par l’État du financement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur l’ensemble de la journée à partir de la rentrée 2024. En outre, au delà de la prise en charge des rémunérations, ce texte permettra une simplification de la gestion des personnels en raison de l’arrêt du cumul de l’emploi entre l’État, chargé du temps scolaire, et les collectivités, chargées du temps périscolaire. La continuité de l’accompagnement des élèves s’en trouvera améliorée. C’est donc d’une avancée importante que nous débattons aujourd’hui ; le vote de votre assemblée devrait acter l’accord définitif entre les deux chambres et permettre la promulgation prochaine de ce texte. Il est de notre devoir collectif de garantir à tous les jeunes, quels que soient leurs besoins spécifiques, une société accueillante qui sache s’adapter. C’est pourquoi, au delà de ce texte qui concerne tout le Gouvernement, l’éducation nationale travaille d’ores et déjà à une évolution de la formation des enseignants et de tous ses personnels.

Le soutien aux personnes en situation de handicap est au cœur de l’action du Gouvernement et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’école. Je me félicite que nous puissions nous rassembler sur un tel sujet. Nous le savons, le chemin est encore long vers cette école pour tous que nous voulons et que nous devons à nos concitoyens, mais nous avançons dans la bonne direction. Permettez moi de saluer Cédric Vial, qui est à l’origine de ce texte, pour son engagement important sur ce sujet

c’est toujours un moment particulier que celui où l’on voit une proposition de loi sénatoriale aboutir. Le texte de notre collègue Cédric Vial, dont je salue de nouveau l’engagement, est de cette espèce ; il nous rassemble au delà de nos clivages politiques. Cette initiative apporte une réponse à des milliers d’enfants, à leurs familles et aux accompagnants d’élèves en situation de handicap. Depuis près de vingt ans, les gouvernements successifs ont mis en place une politique volontariste d’inclusion scolaire. Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a quadruplé : il est passé de 118 000 en 2006 à 478 000 à la rentrée 2023. Cette hausse pose mécaniquement la question de l’accompagnement de ces enfants sur le temps méridien. Or la décision du Conseil d’État du 20 novembre 2020 a dégagé l’éducation nationale de toute responsabilité dans la prise en charge financière des AESH en dehors du temps scolaire. À rebours de la pratique qui existait jusqu’alors, elle a causé un séisme dans les modalités d’accompagnement des élèves concernés sur le temps méridien. Depuis plus de trois ans, les familles et les accompagnants d’élèves en situation de handicap, les précieux AESH, sont confrontés à de nombreuses incertitudes et difficultés. Surtout, cette décision a ouvert la voie à des inégalités de traitement entre les élèves. À l’Assemblée nationale, Mme Belloubet a indiqué que le ministère de l’éducation nationale continuait d’assurer la prise en charge financière sur le temps méridien de 60 % des élèves en situation de handicap. Qu’en est il alors des 40 % restants ?

J’avais également évoqué, lors de l’examen de ce texte en première lecture, le cas des établissements scolaires privés sous contrat. Les sommes qu’ils perçoivent au titre du forfait scolaire ne peuvent être utilisées au profit du temps périscolaire. Des responsables d’établissements scolaires m’ont expliqué devoir jouer sur la solidarité en faisant appel à des volontaires parmi les parents ou les enseignants retraités. Parfois, des AESH sont présents sans refacturation par leur rectorat, et chacun fait comme si cela était possible. C’est ainsi un bricolage qui est mis en place, et qui fonctionne

Madame la ministre, je me félicite de l’évolution du Gouvernement sur ce sujet : il y a quelques mois encore, il y était plutôt réticent. En première lecture au Sénat, votre collègue Catherine Vautrin, ministre de la santé et des solidarités, « une position de sagesse particulièrement bienveillante » sur ce texte, signalant ainsi un infléchissement de position. Quelques jours plus tard, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé le transfert à l’État de la prise en charge des AESH sur le temps méridien. Cette déclaration a bien entendu été unanimement saluée dans notre hémicycle. Le texte issu de l’Assemblée nationale comporte des modifications mineures, principalement rédactionnelles ou de précision. Aussi la commission de la culture l’a t elle adopté conforme en deuxième lecture. Les députés y ont ajouté deux articles. L’article 3 précise que ce texte entrera en vigueur à la rentrée scolaire de 2024. Il semble en effet opportun de prévoir une entrée en vigueur différée de quelques semaines, afin de procéder aux ajustements juridiques nécessaires dans les contrats des AESH. Madame la ministre, j’appelle votre attention sur la demande de rapport inscrite à l’article 4. Vous connaissez la position traditionnellement réservée du Sénat sur ce sujet. prévu dans ce texte porte notamment sur le nombre d’élèves concernés par un accompagnement sur le temps méridien et sur les notifications non couvertes.

fondée sur l’extrapolation d’un sondage réalisé il y a quelques années. Des informations plus précises sur ces thématiques seront donc les bienvenues et j’ai toute confiance dans les capacités statistiques du ministère pour nous éclairer.

Surtout, elle ne constitue qu’un jalon dans un parcours long visant à améliorer la prise en charge des élèves en situation de handicap à l’école.

neuf autres ne relèvent pas de la compétence du législateur ; madame la ministre, j’espère qu’elles connaîtront le même accueil positif de la part du ministère de l’éducation nationale et qu’il y sera donné suite. Enfin, permettez moi de saisir cette occasion pour vous alerter sur la situation de l’école inclusive, aujourd’hui en souffrance.

En 2023, les trois quarts des enseignants du premier degré déclaraient avoir des difficultés fréquentes ou très fréquentes avec des élèves désignés comme perturbateurs ou à troubles du comportement. Il est urgent d’entendre ce malaise professionnel qui remet en cause le bien être de tous à l’école. En effet, c’est l’ensemble de la classe, l’enseignant et l’élève concerné qui souffrent face aux carences des acteurs institutionnels. Mes chers collègues, dans quelques minutes, nous allons adopter définitivement ce texte. Je souhaite qu’il puisse améliorer dès la rentrée prochaine le quotidien des milliers d’enfants concernés ainsi que celui de leurs familles. Une pierre après l’autre, texte après texte, nous œuvrons au Sénat pour bâtir la promesse républicaine d’une école pour tous. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis pour faire aboutir l’adoption de cette proposition de loi visant à assurer la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne. Cette avancée, qui se concrétisera dès la prochaine rentrée scolaire, nous permettra de retrouver de la clarté dans l’accompagnement de la scolarité des élèves en situation de handicap sur ce temps de pause, et ainsi de revenir aux principes fondateurs de l’inclusion scolaire. Le revirement provoqué par la décision du Conseil d’État du 20 novembre 2020, qui a renvoyé aux collectivités territoriales le financement de l’inclusion sur le temps de pause méridienne, a été source de multiples difficultés et incertitudes pour l’ensemble des acteurs impliqués.

Pour les accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap, ensuite, cette dualité d’employeurs a rendu plus compliquée l’organisation de la journée de travail, au détriment notamment de leur propre temps de pause. et bien sûr, les élèves en situation de handicap ayant des besoins d’accompagnement sur le temps méridien, dont le nombre est estimé entre 20 000 et 25 000, confrontés au risque d’une rupture d’accompagnement entre temps scolaire et temps méridien, ce qui a contraint certaines familles à prendre le relais pendant la pause méridienne, à recourir à des AESH privés, voire à déscolariser leurs enfants.

sur le cadre confus et hétérogène résultant de cette décision et sur la nécessité de réaffirmer, par une évolution législative, le principe de l’égalité d’accès des élèves au service de restauration. Je remercie également la rapporteure de ce texte, Anne Ventalon, pour le travail mené au fil de l’examen de cette proposition de loi, qui a permis de mettre encore davantage en lumière les conséquences délétères de ce changement jurisprudentiel. Nous étions unanimes lors de l’examen de ce texte, en janvier dernier, et nous pouvons constater qu’à l’Assemblée nationale le consensus a également été large pour l’approuver, les évolutions intervenues à l’occasion de la navette étant mineures. Je souhaite toutefois revenir sur l’article 4 introduit à l’Assemblée nationale, qui prévoit la remise d’un rapport visant notamment à indiquer le nombre d’élèves concernés par ces accompagnements pendant la pause méridienne et à dresser un état des lieux des prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées pour le temps scolaire et le temps de pause méridienne. Cet article m’interpelle, car il confirme que, sur le sujet de l’école inclusive, le Gouvernement continue de progresser à tâtons. Nous mettons pourtant en garde depuis plusieurs années sur l’urgence d’une réflexion globale et concertée concernant l’organisation de l’école inclusive, dans un contexte où le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a quadruplé entre 2006 et 2023, et où près de neuf élèves en situation de handicap sur dix sont désormais scolarisés en milieu ordinaire.

un véhicule législatif inadapté, à savoir le projet de loi de finances pour 2024. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs censuré l’article correspondant. Quelle n’a donc pas été notre surprise d’apprendre au détour d’une audition de la ministre de l’éducation nationale par notre commission de la culture que, en dépit de cette censure, les pôles d’appui à la scolarité étaient d’ores et déjà en cours d’expérimentation dans quatre départements ! La représentation nationale doit être associée à toute évolution structurelle de l’école inclusive. J’ajoute que celle ci ne doit pas être pensée dans une logique de rationalisation budgétaire, mais qu’il faut s’attacher à répondre avant tout aux besoins des élèves en situation de handicap.

nous le savons, leur rémunération moyenne s’élevait à 994 euros en janvier 2024, soit une précarité indigne pour le deuxième métier de l’éducation nationale.

La fierté, tel est le sentiment qui m’envahit au moment où je vous parle : la fierté d’avoir fait d’un constat un projet, puis d’en avoir fait un combat, et maintenant une loi. La fierté, ce n’est pas de l’orgueil ; c’est le sentiment que l’on ressent quand on a l’impression d’avoir servi à quelque chose. C’est justement le fait de pouvoir vivre ce genre de moments qui donne du sens à notre engagement et à l’action politique. C’est la possibilité de se sentir utile qui nous incite à poursuivre, en dépit d’un contexte qui n’est pas toujours simple ni engageant. Plus qu’une conclusion, ce moment est un aboutissement : celui d’un travail de plus d’une année, ce qui reste malheureusement, en politique, un temps relativement court. Après avoir soulevé un certain nombre de problèmes auprès du Gouvernement à l’automne 2022, après avoir conduit une mission d’information dont les conclusions ont été rendues le 3 mai 2023, j’ai déposé cette proposition de loi en juillet 2023. Elle deviendra une loi, ce soir, après votre vote que j’espère conforme, pour s’appliquer dès la rentrée scolaire 2024. Permettez moi d’adresser ici quelques remerciements. tout d’abord Laurent Lafon, le président de notre commission, qui m’a suggéré le premier la réalisation de cette mission d’information. Merci à Max Brisson et à Philippe Mouiller, qui m’ont aidé, accompagné et soutenu dans ce travail. Merci à Bruno Retailleau et à Gérard Larcher, qui ont permis, parce qu’ils y croyaient, l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de notre assemblée. Merci à Anne Ventalon,

qui ont voté ce texte à l’unanimité lors de la première lecture au Sénat et dont je ne doute pas qu’ils feront de même ce soir. Merci aussi aux députés, qui ont également voté le texte à l’unanimité, à l’exception notable, tout de même, du groupe de La France insoumise, qui n’a pas osé voter contre, mais qui n’a pas su voter pour. est un aboutissement, mais non une fin. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à cette tribune, cette loi simple permettra de régler des problèmes complexes. Elle était nécessaire, mais elle est loin d’être suffisante. Elle répond à une préconisation de mon rapport sur l’organisation de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Ce rapport en compte dix neuf autres, auxquelles il faudrait ajouter, bien sûr, le travail qui reste à mener sur le statut, la rémunération et les conditions de travail des AESH. Ce soir, j’ai donc une pensée toute particulière pour tous les enfants en situation de handicap scolarisés dans notre pays, qui sont près de 480 000, pour tous les AESH, qui font un beau métier, parfois mal considéré. Ils sont près de 140 000 agents, dont près de 97 % sont des femmes. J’ai aussi une pensée pour toutes les familles concernées, pour les enseignants, les agents de cantine, pour les élus locaux, maires, adjoints aux affaires scolaires ou au handicap, ainsi que pour les chefs d’établissements publics et privés. Nous répondons ce soir à l’une de leurs attentes, mais il reste tant à faire encore pour que l’école inclusive

ils sont plus de 130 000 en France et ils attendaient de notre part, de la part de la représentation nationale, un geste fort de reconnaissance et d’aide ; c’est un premier pas que ce soir nous faisons. L’accompagnement des plus fragiles par l’État est un enjeu majeur, preuve d’une société qui va bien. En effet, offrir un soutien humain et humaniste est un impératif moral et éducatif. La prise de conscience du Gouvernement sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap, bien que Intégrer ces enfants favorise la sensibilisation, la tolérance et le respect mutuel : c’est l’occasion pour tous de mettre en pratique nos valeurs fondamentales d’égalité, de respect et de solidarité.

En effet, cette charge reposait jusqu’à présent sur les collectivités locales, ce qui créait une disparité territoriale selon la volonté politique de chaque collectivité, mais aussi et surtout, madame la ministre, selon leur capacité à financer un tel dispositif avec le peu d’argent que vous voulez bien leur laisser. L’État va enfin prendre ses responsabilités et financer un objectif national, prenant conscience qu’un enfant en situation de handicap a besoin d’un accompagnement total pour être intégré pleinement dans le système scolaire et périscolaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. Je souhaite tout d’abord rendre hommage à l’action déterminante de notre collègue Cédric Vial, auteur de cette proposition de loi qui permet non seulement de tenir compte des réalités de vie des enfants handicapés et de leurs familles, mais aussi de soulager le budget des collectivités territoriales dans le contexte très tendu qui est celui des finances locales. Je n’oublie pas non plus le remarquable travail de fond effectué par notre rapporteure Anne Ventalon, que je tiens à souligner. Comme je le précisais il y a quelques jours lors de la réunion de la commission de la culture, ce sujet a largement préoccupé les élus locaux pendant la campagne des dernières élections sénatoriales. solution soit trouvée au problème du manque de leviers de financement dont ils disposent. Ils sont également très démunis pour répondre à la détresse des familles concernées, même si certaines communes, notamment en Essonne, ont décidé de manière volontariste de prendre en charge financièrement l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de la pause méridienne. Certains établissements scolaires, ceux de l’enseignement privé sous contrat, ont eux aussi dû faire face à un dilemme : trouver les financements nécessaires ou laisser les familles assumer un coût bien trop lourd pour elles. En dépit de ces solutions relevant de la seule initiative des collectivités territoriales ou des établissements d’enseignement, de nombreux enfants handicapés se retrouvent aujourd’hui sans éducateur rémunéré pour les accompagner pendant la pause méridienne. Dans l’urgence, les familles ont dû s’organiser, mettre parfois leur vie professionnelle entre parenthèses, investir un budget considérable dans l’éducation de leurs enfants – situation ô combien insupportable Cette proposition de loi met donc un terme aux difficultés engendrées par une décision du Conseil d’État, certes fondée en droit, mais humainement inacceptable. Nos collègues de l’Assemblée nationale ont souhaité apporter quelques modifications au texte adopté en ces murs en première lecture d’une part, des modifications d’ordre rédactionnel ; d’autre part, l’ajout de deux articles supplémentaires. Les députés ont notamment prévu la remise d’un nouveau rapport. Il est vrai que nous n’avons pas pour habitude, au Sénat, de soutenir ce genre d’initiative. Pourtant, Pourtant, comme cela a été largement dit en commission, il n’est pas utile de prolonger la navette parlementaire : nous voulons permettre l’application de cette loi dès la rentrée prochaine. Les familles ont déjà bien trop attendu et les élus nous demandent d’agir instamment.

pour tous, partout ; cette proposition de loi y participe de manière concrète. Mais, comme je le soulignais lors de mon intervention en première lecture, il nous faudra aussi imaginer l’école inclusive de demain et travailler à des avancées concrètes pour les AESH, dont les conditions d’emploi et de travail éprouvantes, pour ne pas dire indignes, doivent faire l’objet d’une réforme structurelle. Il nous faudra par ailleurs accélérer la prise en charge des élèves qui ne peuvent être scolarisés en milieu ordinaire et prévoir des créations de places dans les établissements médico sociaux, en particulier les

mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier notre collègue Cédric Vial, auteur de cette proposition de loi, et la rapporteure Anne Ventalon. Ce texte est très attendu, car il constitue une réponse concrète à un problème réel.

En novembre 2020, le Conseil d’État a dispensé l’État de la prise en charge des AESH sur le temps périscolaire. Cette décision a provoqué de nombreuses difficultés pour les élèves, leurs familles et les établissements scolaires. Des dizaines d’enfants ont dû être déscolarisés, faute de moyens. Les parents qui embauchent eux mêmes un accompagnant pour la pause méridienne doivent débourser 400 euros par mois ! Le 23 janvier 2024, nous avons adopté cette proposition de loi en première lecture. Elle a pour objet de rétablir l’égalité d’accès à l’éducation en instaurant la prise en charge par l’État des AESH sur le temps méridien.

Ce texte fait consensus. Si nous nous réjouissons tous de l’avancée qu’il représente, je m’interroge sur sa mise en œuvre. Madame la ministre, vous avez indiqué que cette mesure, chiffrée à 31 millions d’euros, nécessiterait entre 2 000 et 3 000 à la rentrée prochaine. Cela représente un véritable défi compte tenu de la pénurie de professionnels : les difficultés de recrutement persistent et persisteront. Un exemple illustre la détresse des familles : le 29 janvier 2024, des parents d’élèves postaient sur le site une petite annonce pour recruter deux AESH. Ce métier, exercé à 93 % par des femmes, souffre d’un déficit d’attractivité.

Pénurie de professionnels, crise d’attractivité, formation et rémunération sont autant de freins au recrutement. Madame la ministre, comment résoudre cette équation ? D’un côté, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire explose – il est passé de 134 000 à 430 000 en près de vingt ans. ans. De l’autre, nous peinons à recruter de nouveaux personnels. Autre constat : chaque année, le nombre d’élèves en situation de handicap augmente de 6 %, alors que le nombre de notifications d’accompagnement humain augmente, lui, Grâce à la loi Vial, accompagner un enfant en situation de handicap signifiera désormais l’accompagner sur les temps scolaire et méridien. Ce texte est une première avancée qui en appelle d’autres. L’accompagnement d’un enfant doit s’entendre sur l’intégralité d’une journée

privilégiés avec le collectif. La proposition de loi de notre collègue Cédric Vial constitue un pas supplémentaire sur le chemin de l’école inclusive, et le groupe Union Centriste se réjouit de la voir aboutir

d’inclusion des élèves en situation de handicap à l’école. L’école inclusive vise en effet à instaurer un peu d’égalité en offrant à ces enfants, dont le besoin d’accompagnement est particulier, des conditions de scolarisation et de sociabilité plus proches de celles des autres enfants. En cela, l’inscription de l’idée d’école inclusive dans la loi est un progrès.

Leur formation et leur rémunération restent très insuffisantes ; la précarité demeure la norme en raison de temps partiels souvent imposés. Il est tout simplement indigne que l’État prévoie de telles conditions de recrutement. situation, beaucoup de collectivités territoriales se sont organisées pour pallier les limites du cadre imposé par le ministère de l’éducation nationale. Comptant parmi les zones d’ombre de la législation actuelle, la question de la prise en charge des élèves en situation de handicap la pause méridienne a fait l’objet d’un long bras de fer entre les collectivités et les ministères. Dans de nombreuses écoles, les accompagnants n’étaient pas rémunérés pour aider ces élèves au moment du déjeuner. je suis fière que de nombreuses collectivités, notamment écologistes, aient anticipé le problème et pris le sujet à bras le corps sans attendre de solution législative. Je remercie notre collègue Cédric Vial de proposer les présentes modifications, qui apporteront des solutions concrètes aux élus de terrain. Bien que des améliorations soient encore souhaitables, nous voulons aujourd’hui une adoption conforme du texte ; c’est pourquoi nous n’avons pas déposé d’amendement. Pourrons nous collectivement faire preuve d’autant de lucidité et de pragmatisme lorsque nous aborderons la question des inégalités de financement, par exemple, entre l’école publique et les écoles privées ?

je pense bien sûr au « choc des savoirs ». Je redoute que, hors cadre légal et sans anticipation des besoins nécessaires à sa mise en œuvre, ce projet ne donne lieu à des complications plus importantes encore que celles qui ont entouré

Merci

le système scolaire français tend à se transformer pour permettre à tous les élèves, notamment à ceux qui sont en situation de handicap, d’accéder à l’école et aux apprentissages. Dit autrement, l’école française a accepté de se repenser, afin de s’adapter aux besoins de tous les élèves, y compris de ceux qui, jusqu’alors, étaient exclus d’une scolarisation que je qualifierai d’ordinaire.

Pourtant, avec cette proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, l’école inclusive est encore devant nous.

En effet, pour parvenir à une bonne pratique de l’inclusion, il faut une école de qualité et de réussite pour toutes et tous. Or force est de constater qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

que nous portions aussi un regard critique sur l’organisation même de notre système éducatif, balloté sans cesse entre inclusion affirmée, d’un côté, et tendance à la sélection des élèves, de l’autre. Le système éducatif français devrait, par une démocratisation de l’accès aux savoirs, offrir à l’ensemble des élèves les mêmes chances de développer leur potentiel.

mais elle tend à régler une partie de la problématique de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Préciser que cette disposition doit entrer en vigueur dès la rentrée 2024 constitue aussi une précision utile.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis une seconde fois en séance publique pour évoquer la prise en charge par l’État de l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps méridien. Vous remarquerez, mes chers collègues, que j’ai sciemment employé le terme « seconde » et n’ai pas parlé de « deuxième lecture ». Ce n’est pas une erreur, bien au contraire : j’espère sincèrement que cette lecture sera bel et bien la dernière, grâce à un vote conforme de notre assemblée,

Nous savons tous qu’il y a urgence à rappeler ce que doit la solidarité nationale aux 478 000 élèves en situation de handicap et à leurs familles, ainsi qu’aux 132 000 personnels qui les accompagnent. Permettez moi d’ailleurs de saluer l’action courageuse de ces contractuels, femmes et hommes, qui travaillent auprès des enfants et de leurs parents. Cher Cédric Vial, je vous remercie sincèrement de votre heureuse initiative. Elle renoue avec l’esprit de la loi de 2005, qui consacrait l’égalité des chances et entérinait le passage d’une obligation éducative à une obligation scolaire dont l’État devait supporter la charge sur le plan tant financier qu’humain. Depuis Depuis le fameux arrêt du Conseil d’État du 20 novembre 2020, nous avons pu observer que cette mission, ô combien indispensable, pouvait pâtir d’une application inégale sur le territoire national.

la charge financière supplémentaire qui était imposée aux collectivités territoriales, alors que les budgets de celles ci sont de plus en plus contraints., ensuite, la dégradation des conditions de travail des accompagnants d’élèves en situation de handicap due à la réorganisation de leurs emplois du temps et aux multiples contrats liés à ce choix.,

pense notamment au décalage persistant entre l’augmentation des moyens humains et financiers et le nombre croissant d’enfants en situation de handicap demandant à être scolarisés.

Ces sujets n’entrent pas dans le périmètre de cette proposition de loi, je le sais pertinemment. Néanmoins, nous ne devons pas les négliger, et il nous appartient de les aborder sereinement, dans un esprit constructif et volontariste. C’est notre

de ce texte s’inscrit par ailleurs dans la logique d’une volonté commune du Président de la République et du Premier ministre de voir l’État financer l’accompagnement des enfants en situation de handicap pendant leur pause déjeuner.

En effet, dès lors que la prise en charge des AESH durant le temps méridien n’est plus assurée ou qu’un élève est accompagné par un AESH différent au cours des temps scolaire et méridien, il y a rupture dans la continuité de l’accompagnement de ces enfants, qui est pourtant essentielle

des parents embauchent directement des AESH, qui, en plus de représenter une dépense significative pour ces familles, et sans remettre en cause leurs compétences, ne sont pas soumis aux contrôles habituellement réalisés par l’éducation nationale.

Nous ne connaissons que trop bien les situations de précarité auxquels ces personnels peuvent faire face. Elles ne seront malheureusement pas toutes résolues par le texte, mais nous saluons cette avancée.

lequel celui ci a jugé que la compétence de l’État en matière de prise en charge des situations de handicap ne devait porter que sur le temps scolaire.

Il permettra de rétablir une forme de solidarité nationale, afin d’accompagner au mieux les élèves en situation de handicap au sein de notre école. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de cette

On sait combien cette clarification était nécessaire depuis l’arrêt du Conseil d’État du 20 novembre 2020, qui avait plongé les communes dans un grand embarras. Pour avoir été pendant vingt ans adjointe au maire déléguée à l’éducation dans ma commune d’Asnières sur Seine, j’ai pu mesurer, à chaque rentrée scolaire, l’ineptie d’une organisation conduisant les AESH à avoir deux employeurs, l’éducation nationale et la collectivité territoriale, une source de complexité kafkaïenne contribuant au manque d’attractivité du métier.

situation, combien d’élus sont désemparés par la détresse de familles qui attendent, à juste titre, que les pouvoirs publics offrent une vraie prise en charge de leur enfant ? Combien d’enseignants ont des problèmes avec leur classe, parce qu’un enfant en difficulté n’est pas accompagné ?

La professionnalisation amorcée par le décret du 13 juillet 2023, avec la possibilité d’accéder à un CDI après un CDD de trois ans et la revalorisation de la grille indiciaire, n’a pas mis fin aux recrutements à temps incomplet.

tous les élèves ayant des besoins spécifiques. Je sais qu’ils y sont attachés. Espérons aussi qu’elle mettra un terme à la pratique de la mutualisation des AESH par les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) et à leur affectation en fonction de l’offre disponible et non, toujours, des besoins de l’enfant.

le temps méridien proprement dit, l’accueil du soir, qui comprend les études surveillées, et les activités culturelles et sportives. Il faudra y remédier. Pour finir, je me réjouis que, en cas d’adoption conforme, cette mesure soit applicable dès la rentrée 2024. Beaucoup reste à faire pour une école vraiment inclusive, je compte bien continuer à y prendre ma part, ici, au Sénat, où le projet d’une société plus inclusive a toujours été une priorité. La discussion